La séance est reprise nous reprenons la discussion du projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023 dans le Sénat et saisi en application de l'article 47 tirer un. Alinéa 2 de la Constitution dans la discussion des articles nous sommes parvenus à l'amendement numéro 2625 rectifié au sein de l'Arctique. Le liminaire. Et nous reprenons donc la discussion avec 6 amendement faisant l'objet d'une discussion commune. Nous commençons donc par le 2625 rectifié. C'est madame Lubin qui le présente. Merci madame la présidente. Cet amendement par cet amendement. Nous souhaitons supprimer toute référence. Au Au projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 car il n'a pas été adopté et promulgué. Et donc. Il nous paraît peu judicieux, voire même un sincère de se référer à ce projet. Dans cet article. Liminaire voilà. Nous nous posons. Des questions par rapport à la constitutionnalité de ce PLFSS. Rectificatif. Et donc la sincérité des débats.

Merci madame la présidente. Alors. Fin 2022, l'Assemblée nationale a rejeté le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 en première lecture.

Il est donc. Tout à fait surprenant pour. Pas dire plus de retrouver ici cité ce projet de texte qui a donc n'été n'ont été adopté par l'Assemblée nationale et qui est donc. Dépourvu d'existence légale, il est vrai que ça a été adopté par le Sénat qui en a profité au passage pour supprimer plus de 100.000 fonctionnaires. Donc. Cet amendement donc supprime cette référence à ce qui reste quand même ce projet de loi. Merci.

Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes, mes chers collègues. Le projet de loi de programmation a été rejeté par le Parlement en commission mixte paritaire à pour été rejeté par l'Assemblée nationale et après avoir été substantiellement modifié et durci par la droite sénatoriale. D'ailleurs, comme on va rester plusieurs jours je vous si messieurs les miss, vous pouvez m'aider à, à voir quel est l'effet vous rappelez l'amendement de la droite qui proposait 150.000 fonctionnaires en moins quelles conséquences ça aurait sur le financement de la sécurité sociale et des retraites, je ferme la parenthèse. Mais c'est un élément important. Le Parlement a fermé la porte à vos projets de loi ça revient par la fenêtre et vous avez décidé de vous hanter. Es dans le mépris du Parmelan Parlement en imposant une vision que je qualifierais de rigoriste des finances publiques. Votre contraction des dépenses publiques en volume, c'est du jamais vu depuis 2005. Depuis que la France se dote d'une programmation pluriannuelle. Je vous donne les chiffres qui nous sont communs d'ailleurs 1,9% de croissance en moyenne pour la première. 0 7 % de croissance en moyenne pour la seconde. 1% de croissance pour la troisième et une baisse de moins 0 4 % pour la présente loi de programmation 2002 23 2027. C'est du jamais vu. Et la droite et sénatoriales estimait mes collègues des des. Je vous ai beaucoup écouté. Pendant la loi de finances que ça faisait pas le compte. Donc je regarde ce que dit le Haut conseil des finances et ça revient au débat qu'on a eues sur l'article liminaire pourquoi vous nous donnez pas les éléments du Conseil d'État parce qu'on a quand même des éléments qui prouvent quand même qu'il a des doutes à avoir, je cite au Conseil des finances publiques. Dernière avis le gouvernement fait l'hypothèse que l'impact d'un ensemble de réformes. Revenu de Solidarité Active, retraites, assurance chômage apprentissage ferait plus que compenser le Net ralentissement de la population active projeté par l'Insee. Comme il l'avait lancé dans son avis sur le programme de stabilité, le Haut Conseil considère que l'impact de ces réformes sur lesquelles le gouvernement n'a pas fourni

Je suis là. C'était un amendement de repli que nous vous proposons afin de supprimer la référence dans le tableau au projet de loi de programmation des finances publiques qui n'a pas été adopté par le gouvernement. Donc toujours la question de l'insincérité. Que j'ai développé tout à l'heure. Et le 2626 26 6. Alors l'article liminaire du présent. Projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale établit la prévision de déficit public à 5% du PIB en 2023, dont 4% pour le seul déficit structurel. Le déficit structurel correspond au solde public des des effets Directs du cycle économique ainsi que des événements exceptionnels et temporaires. La notion de déficit structurel donne lieu à de nombreux débats méthodologique, puisqu'elle repose sur le concept de croissance potentielle qui est par définition non observables donc non mesurable, en effet, la croissance potentielle et celle qu'aurait l'économie si tous les facteurs de production pouvait être pleinement activées. De ce point de vue l'utilisation d'une méthode de calcul constante au fil du temps permet d'établir des comparaisons d'une année sur l'autre, c'est le calcul auquel procède chaque année, la Commission européenne qui. De composante structurelle et conjoncturelle du déficit de chaque pays et ce, avec la même méthode appliquée dans tous les pays. Dans ses dernières prévisions publiées en octobre 2022. La Commission européenne prévoit des hypothèses supérieure à celle du gouvernement, avec un déficit public de 5,3% du PIB, dont 4,9% de déficit structurel. Le présent amendement vise donc à corriger le niveau du déficit public ainsi que la part structurelle de ce déficit pour les rendre conformes à ceux calculés par la Commission européenne. Monsieur Bocquet. de dealers, de peur comme si contrôler l'action du gouvernement et ses prévisions économiques outrepasser le rôle des oppositions Parlement je vais le citer. Je ne veux pas que certains jouent avec les peurs des Français en disant, récession, chômage vague de faillites, ça ne correspond pas à la réalité et je crois qu'en politique, il est bon de revenir à la réalité et de garder son sang-froid. Fin de citation. Revenir à la réalité impose de se mettre d'accord sur les faits. Est-ce la réalité que les radiations atteignent un record sans précédent en novembre 2022 avec 5058 1100 radié, une première depuis 1996, date du début de recensement de cette statistique. que là il a, que les radiations représente 9,7% des sorties au dernier trimestre de l'an dernier. À manier les arguments autour de la responsabilité en politique à tort et à travers, on finit par s'exposer soi-même et son gouvernement un risque de manque de rigueur et donc être pris à défaut si ce n'est de mensonges, mais de subjectivité démesuré, une forme d'irresponsabilité en somme. Lorsque nous Majoro ont dans cet amendement, le déficit structurel c'est bien parce qu'il y a une intention de vous alerter sur le fait que vos estimations ne sont pas juste et que dès lors, vous ne tiendrait pas les objectifs que vous vous assignez bien sûr, nous ne les partageons pas alors que le déficit structurel et mesurée à moins 4, 9, 9 points par la Commission européenne pour notre pays en 2023. La majorité sénatoriale projeté lors de la loi de programmation une ambition fondée sur, moins 3,6 points de déficit structurel, c'est bien une différence d'approche qui nous oppose cette différence a des conséquences budgétaires extrêmement importante car nos 1000 auront d'autant la part conjoncturelle imputable au déficit public, c'est-à-dire aux mesures temporaires. Les mêmes mesures, dans lesquels le Sénat voulait trouver sa voie de passage pour justifier une austérité plus important. Merci, cher collègue, la parole est à la Commission pour avis sur ces six amendements madame la rapporteure. Oui merci madame la présidente. Oui alors concernant tous ces amendements les premiers concerne en fait la non référence à la loi de programmation des finances publiques. C'est une obligation toute toute article liminaire d'une loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale. Alors faute d'adoption parce que certains évoquent effectivement la non-adoption d'une telle loi. La référence au projet de loi de programmation et la moins mauvaise solution même si cela pourrait poser une difficulté à la longue pour d'autres, vous proposez de rajouter une colonne ou d'en enlever une, là c'est quelque chose d'impossible. Donc c'est un avis défavorable. Merci, monsieur le Ministre avis du gouvernement. Merci madame la présidente. D'abord je vous remercie monsieur Savoldelli. Puisque vous avez dit que le projet de loi de programmation des finances publiques présentées par le gouvernement. Contient l'effort de maîtrise de la dépense publique. Le plus fort depuis 20 ans. Et c'est ce que je me suis évertué à essayer de convaincre la majorité sénatoriale. On a eu de longues discussions avec. Jean-François Husson, sur le sujet avec Bruno Retailleau. Oui, merci Monsieur Salvodelli d'insister sur le fait que la LPFP que nous avons proposé et l'effort historique en matière de maîtrise de la dépense publique, en tout cas depuis 20 ou 30 ans peut-être que vous participerez à convaincre de notre ambition sur sur ce sujet-là. Ensuite, je voulais vous dire que vous vous prenez dans la vie du HCSP ce qui vous arrange parce que il est écrit noir sur blanc dans la vie du HCSP. Que les prévisions d'estimation du gouvernement sur l'impact de la réforme des retraites sont, je cite, réaliste. Ensuite vous proposez dans ces amendements. Plusieurs choses, d'abord, certains proposent.

vous dénoncez vous-même le sentiment que vous pouvez avoir qu'on répondrait à une forme de ces mêmes terme diktats qui est souvent employé et cetera de la Commission européenne, là vous proposer des amendements qui disent parce que la Commission européenne fait une prévision de déficit qui est différente que de celle du Parlement et du gouvernement, il faut immédiatement ajusté mais heureusement qu'il y a un parlement et un gouvernement que c'est pas la Commission européenne qui seul décide de changer nos prévisions, déficit pour l'année 2023 et souvent il y a eu des prévisions et on a vu d'ailleurs dans ce qui s'est réalisé qu'on était plus proche de ce qui avait été prévu par le gouvernement et par le Parlement. Ensuite vous proposer pour certains d'entre vous, enfin pour l'intégralité des amendements de supprimer la référence au projet de loi de programmation des finances publiques sous prétexte que celui-ci n'ayant pas été adoptée, cela rendrait je cite certains d'entre vous hein. Sincère, le texte puisqu'il se réfère à un projet de loi qui n'a pas été adopté par le Parlement. C'est précisément ce qui s'est passé dans les textes financiers à l'Automne dans les textes financiers à l'Automne qui ont été adopté je le rappelle ici. Article liminaire référence au projet de loi de programmation des finances publiques qui à l'époque non plus n'avait pas été adopté. Ça a été jugé par le Conseil constitutionnel, décision du Conseil constitutionnel du 22 décembre 2022 dans son considérant numéro 23 je crois. Que dit le Conseil constitutionnel. Le projet de loi de finances fait référence au projet de loi de programmation des finances publiques n'a pas encore été adoptée, alors que la loi de finances est adopté. Mais ça n'est en aucun cas une méconnaissance de la loi organique et une loi de finances, une loi de financement de la Sécurité sociale un PLFR un PLFRSS peut tout à fait faire référence, un projet de loi de programmation des finances publiques non encore adoptés donc ça fait tomber vos arguments selon lesquels ce serait. Un pas respecter la loi organique ou ce serait rendre un ce texte donc avis défavorable pour toutes ces raisons. Merci monsieur le ministre. Explications de vote, monsieur le président.

m'a semblé et m'a semblé que dans ses préliminaires. Monsieur le Ministre des comptes publics. Vous avez évoqué régulièrement sur des propositions qui étaient faites par mes collègues. Que finalement. La baisse de l'impôt sur les sociétés s'était traduit par une augmentation du produit. Alors j'ai quand même été regardé de près quoi c'est toujours intéressant de regarder de près et j'ai vu que le produit finalement de l'impôt, il était de finalement depuis 2006 à peu près hors évidemment, période de crise. 2008 2009 2010. Vous le comprendrez mais on retrouve à peu près 50 milliards et on est évidemment maintenant 50 milliards en 2006 et c'est les chiffres que j'aime et que c'est votre ministère vous savez. Oui bon alors même 60 milliards. Eh bien non, non l'année dernière on était à 48 milliards. Bon voilà, je voudrais vous le rappeler c'est du juste pour vous dire, en 2021 on était à 40 milliards à 2021. Et donc je ne sais pas vous dire simplement que quand on a baissé le taux pour l'instant ça s'est pas traduit par une augmentation sensible de la recette. D'autre part, on est sur des impôts qui sont extrêmement fluctuants, vous le savez parce que d'une année à l'autre et qu'il se calcule. Il se modifie. Parce que c'est, ils sont très compliquées à calculer et en particulier ça joue beaucoup sur les acomptes et la période d'acompte fait que il y a un suivi qui est un peu. Pas très linéaire des choses donc en tout cas, Monsieur le Ministre. Je vous encourage pas à développer cet argumentaire que d'ailleurs France stratégique et le le service placé auprès du Premier Ministre ne confirme pas pour l'instant s'il ne le confirme pas pour l'instant, soyez prudents. Merci. Si cher collègue, Monsieur Féraud pour explication de vote. Merci madame la présidente. Tendu l'argumentation du ministre-tout à l'heure mais enfin regarder la situation dans laquelle nous sommes, nous sommes finalement en train de discuter d'un texte. Qui n'a pas été voté par l'Assemblée nationale. Et qui êtes argumenté dans son article liminaire sur un texte qui n'a pas non plus été voté par l'Assemblée nationale, on peut faire du juridisme mais il y a un problème de légitimité démocratique dans notre discussion et dans ce projet de loi le gouvernement aurait d'ailleurs pu faire adopter la loi de programmation des finances publiques par l'article 49.3 à l'Assemblée nationale, il n'a même pas estimé que cela était nécessaire, donc nous avons là aujourd'hui un texte qui s'appuie sur un projet de loi non adopté, enfin plus exactement, il a été adopté ici au Sénat, mais dans une version qui ne convient même pas au gouvernement, une forme d'honnêteté intellectuelle serait au moins de supprimer cette référence au projet de loi de de programmation des finances publiques dans ce PLFSS en ordre, de matière de en matière juridique et que chacun reconnaisse qu'il y a un problème de légitimité démocratique dans notre discussion aujourd'hui. Merci monsieur Faure. Il n'y a plus d'explications de vote, je mets Monsieur Bruillet monsieur à Monsieur Bruillet. Merci madame la présidente. Oui, une explication de vote parce que comme vient de l'expliquer Rémi Féraud. Je vous avoue que pour un jeune sénateur comme je suis, c'est assez étonnant et troublant de. Ah récent oui et c'est c'est plus juste que je suis assez d'accord c'est c'est plus juste de dire récent sénateur. Et donc pour un sénateur, récemment installé. J'ai entendu avec bonheur. L'ensemble de ces bancs défendre souvent face au gouvernement. La sincérité des débats et l'exigence du travail bien fait pour le Sénat, et dans ce texte nous nous appuyons donc sur des des des orientations qui n'ont pas été validé. Celle du projet de loi de programmation. Moi je ne sais d'ailleurs pas qu'elles sont pas ce qu'elles sont puisque ici dans cette amitié que nous avons voté la suppression de 120.000 emplois de fonctionnaires. Enfin, nous vous avez voté chers collègues à droite la suppression de 120.000 emplois de fonctionnaires et je ne les retrouve pas dans les tableaux c'est 120.000 emplois supprimés. Je ne n'retrouve pas dans les tableaux et comme ensuite le texte n'a pas été adopté. Je ne sais pas quel est le texte qui reste en course mais 2ème remarque vous n'acceptez pas, Monsieur le Ministre Dussopt de communiquer aux parlementaires la note de synthèse du Conseil d'État. Certains de mes collègues vont penser que je suis redondant. C'est pas faux. C'est pas faux mais je m'attendais à ce que sur vos bancs aussi on demande cette note de synthèse du Conseil d'État. Ça fait partie de la bonne information des parlementaires et de la sincérité des débats et entendre un ministre nous dire que de toute façon c'est connu, il suffit de lire les journaux ne me paraît pas respectueux du travail parlementaire. Merci la parole à monsieur Savoldelli et en. Le tiendra par la prise de parole de monsieur le Ministre. Merci madame la présidente. Bonsoir. Sur les ministres, mes chers collègues, monsieur Attal, je viens de retrouver vos propos à l'Assemblée nationale. Dixit. Je vous cite me fait pas perte de temps. Il y a toujours un projet de loi de programmation des finances publiques ne vous en déplaise. Et ce n'est pas très respectueux du Sénat que de considérer que quand le Sénat vote un texte cela signifie rien. Hé ben ici on est au Sénat. Donc le Sénat il a modifié le projet de loi et il a durci dedans il y avait la suppression des 120.000 fonctionnaires qui n'a pas été retenue et il y avait d'autres aspects. Vous en tenez pas compte dans les propositions, vous nous faites là. Ici on au Sénat et les sénateurs ont rejeté en CMP vous en tenez pas compte non plus. Alors oui a un projet de loi de programmation des finances publiques. Je sais pas où il est. On en a on n'y a pas accès. Si on n'y a pas droit. On y a pas droit à qu'on soit de la majorité ou de l'opposition n'y a pas droit je ai pas dans quel tiroir il est mis et j'ai regardé comment vous fondez vos décisions sur comment vous interprétez la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2022 qui aurait, je cite son considérant 23 et là je le cite, Monsieur le Ministre. Je cite en l'espèce. Le tableau de synthèse de l'Arctique liminaire de la loi de finances pour les 2023 reprend les prévisions présentées dans le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 2027. Si ce projet de loi de programmation qui a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, le même jour que le projet de loi de finances n'a pas été adopté avant l'adoption de la loi de finances pour 2023, il ne résulte de cette circonstance aucune connaissance de l'article 1er rage de la loi organique du premier août 2001. Du principe de clarté. Et du principe de sincérité du débat parlementaire, donc les choses sont claires. On travaille dans quelles conditions ici. Avec quel respect des travaux parlementaires. Franchement et puis tout à l'heure sur la question, vous choisissez sénateur Savoldelli un passage de ce que dit le Haut Conseil ça vous voyez ça. On choisit pas moi je choisis pas ce que sont les avis du Conseil d'État

D'abord je vous rassurer joue moi je crois profondément que la jeunesse est un état d'esprit et j'ai appris tout à l'heure par Madame Rossignol que j'étais un vieux thatchérien donc. Ça veut dire qu'il pouvait être un jeune sénateur. Ensuite. ensuite je veux vous vous préciser puisque c'est une question que vous avez posé de clarté. C'est bien par rapport au projet de loi initial déposé par le gouvernement sur la loi de programmation des finances publiques que se fonde cet article liminaire parce que le texte est encore dans la navette parlementaire. Donc les écarts qui sont mesurées dans l'article liminaire, c'est par rapport au projet de loi initial. Hé oui monsieur Savoldelli vous avez lu vous-même le considérant 23 de la décision du 29 décembre 2022 du Conseil constitutionnel qui dit très clairement qu'un texte financier peut tout à fait se référer à un projet de loi de programmation des finances publiques non encore adoptée sans que ça n'ait aucun impact sur la sincérité des débats et que, sans ça n'ai aucun a aucun impact sur le respect, la loi organique mais c'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil constitutionnel. enfin on le respecte tous je crois et enfin pour répondre à Monsieur rénale. L'an dernier recettes d'impôt sur les sociétés historiques, 62 milliards d'euros en 2006, l'année que vous avez pris en pris en référence, je crois que c'était entre. Combien. 45. En 2006, le tout à l'époque était à 33% d'avait 45 aujourd'hui, le taux est à 25%, on a 62, donc c'est plutôt positif et sur France Stratégie. Je veux pas allonger les débats. On n'est pas en PLF évidemment mais France stratégie rapport très intéressant sur le prélèvement forfaitaire unique la flat tax. Ils disent quoi que la flat tax prélèvement forfaitaire unique s'est financer parce que le fait qu'on ait baissé les impôts a fait que l'activité économique s'est développée que les recettes supplémentaires ont compensé la baisse du tout, donc c'est plutôt positif aussi du point de vue de France Stratégie. Merci monsieur le ministre, hein. J'ai été saisi. D'une demande de scrutin public par le groupe socialiste, écologiste et républicain. Sur les trois amendements identiques, 2625 3402 3813. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable. L'avis du Gouvernement défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. Le résultat votants 343 exprimés, 343 pour 91 contre 252. Ces trois amendements ne sont pas adoptés. Le 2627 a reçu 2 avis favorable même vote.

Qui est contre. La. Qui s'abstient. Il n'est pas z'adopté 3806 2 avis défavorables qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas Z opté 4478. Qui le défend. Madame. Madame Assassi Madame Bruna il est défendu.

Madame Assassi Nous considérons que. L'expression d'être au sens de Maastricht aura invisibiliser le caractère contraignant d'un traité européen en l'occurrence celui de Maastricht qui, par la coordination de politique économique, c'est-à-dire l'article 121 et la formule lapidaire de l'artiste sur je cite les États membres et évite les déficits excessifs consacrent joue des institutions européennes. À l'instar des décisions nationales en matière de dépenses publiques. Je vous l'ai dit, ça va bien se passer. Donc cette réforme des retraites. Il convient de la rappeler et de le rappeler, émane d'une volonté européenne de réduction de la dépense publique dont cet amendement permet de ne pas omettre la jeunesse si le sens de cet amendement. Merci madame la présidente, avis de la commission sur le 4478. Oui. Madame la présidente Assassi. La vie de la. La commission est défavorable. Là moi je reconnais votre.

Je pense que en fait le sens il est là à Maastricht, tout le monde comprend et donc est-ce que ça vaut le coup finalement de prolonger la navette sur cet article, je ne le pense pas. À ce. Merci madame la va la rapporteure. Monsieur le Ministre défavorable Monsieur Laurent. D'abord Madame Rossignol ensuite s'il faut qu'on maintenir dans tous les textes budgétaires cette formule, la dette au sens de Maastricht, les critères de Maastricht, tout le monde les connaît, ils ont volé en éclats avec la pandémie, il y a plus aucun pays européen qui les respecte. Donc les critères de Maastricht, ne sont pas respectés en Europe actuellement. Plus personne ne parle de la règle des 3% et d'ailleurs le pacte budgétaire est suspendu et personne à ma connaissance ne connaît les règles futur puisqu'elles sont en négociation. À moins que le gouvernement les ait décidé tout seul sans ses partenaires européens. Donc pour le moment, les règles de la dette au sens de Maastricht, on ne sait pas ce que ça veut dire. Par ailleurs, nous savons aujourd'hui que le calcul sur lequel reposait ça était parfaitement artificielle je vous prendre des chiffres. La dette publique au sens de Maastricht comme vous dit elle s'élève en 2021 à 112% et demi du PIB. Mais au sens de l'Insee les mêmes chiffres, c'est 101 de du PIB et au sens de d'Eurostat et de l'OCDE. Ces 87% du PIB. Donc en fait il y a débat sur ces critères, vous continuez de les utiliser comme un dogme qu'ils étaient au départ alors qu'ils n'ont plus de sens aujourd'hui surtout dans la situation dans laquelle nous sommes. Donc c'est ça la question que nous posons. Vous continuez d'agiter ce dogme pour justifier la compression des dépenses en faveur des retraites alors qu'en vérité ces règles elles ont volé en éclats aujourd'hui. Merci monsieur le président, madame la prise entre Signol. Je pense que certains d'entre nous peut être beaucoup voteront cet amendement mais je voulais juste revenir sur le l'argument qui avait été donné par la rapporteure qui disait qu'il ne fallait pas changer d'être de Maastricht par du traité de Maastricht parce que ça risquait de ralentir inutilement la navette et j'ai un doute sur la je prends quand j'ai pas tout compris en fait sur ce qui se passe en ce moment, dès lors qu'il n'y a pas eu à l'Assemblée nationale d'adoption de ce texte. Quelle navette pourrait être ralentie par le fait que nous votons un amendement et je voudrais savoir si cet amendement ralentirait plus la navette que les amendements que vous allez proposer tout à l'heure à l'article 2 sur les régimes spéciaux. Alors que l'article 2 a été rejeté à l'Assemblée. Qui risque aussi de retarder la navette donc qu'est-ce que la navette vient faire un Maastricht dans cet article là je n'ai pas compris mais on votera l'amendement quand même parce que d'amendement. J'ai compris. Merci, cher collègue, la parole est à Madame Lienemann. Oui, chers collègues, le terme de dettes Maastricht yen n'a pas de sens. Je vous rappelle que le traité de Maastricht. Ne fais fixait pas à des critères durables. C'était des critères de convergence. Dont la fin de vie de ces critères obligatoires était le passage à l'euro. Et c'est le traité d'Amsterdam. Qui redéfinit le cadre du pacte de stabilité. Donc les critères de dettes. Ne sont pas définies dans le tri, critères de Maastricht, puisqu'ils étaient caducs au moment du passage à l'euro mais ceux d'Amsterdam, ce n'est pas neutre politiquement. Car tous ceux qui ont voté Maastricht n'ont pas nécessairement voté le traité d'Amsterdam. Une chose était de converger. Une autre était de mètres dans le dogme des traités des critères macro-économique qui devrait relever de l'arbitrage politique. Mais je voudrais dire un autre point, c'est que un des critères. Qui n'est jamais soulevé. Et qui devrait pourtant être soulevée par la France vis-à-vis de l'Allemagne. C'est le critère de de balance. De de balance commerciale excessive. Il était prévu dans les traités. Que si un pays de l'Union. Avait une balance commerciale excessivement forte. Au regard de la moyenne. Il devait prendre des mesures de relance intérieure pour justement rééquilibrer la donne, notamment en matière d'échanges industriels. J'observe que la France n'a jamais eu le courage de demander le respect de ces critères. En tout cas ils ne sont pas de Maastricht mais du traité d'Amsterdam. Merci cher collègue hein. Je vais mettre aux voix l'amendement 4478 qui a reçu 2 avis défavorables. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté le 3793. Madame brûle. Merci madame la présidente. Il est proposé avec cet article dans. C'est une ligne qui précise les objectifs réels de cette réforme a savoir contenir la croissance des dépenses de Sécurité sociale et de retraite, à 0,6%, afin de se conformer aux engagements pris auprès de la Commission européenne de maintenir une croissance des dépenses publiques à 0 6 %. Je crois que dans cet article. Nous voyons. À nouveau, je serais tenté de dire. Quel est le véritable projet du gouvernement, il ne s'agit pas seulement de faire travailler plus longtemps les Françaises et les Français pour soi-disant sauver notre système de retraite par répartition, ni d'améliorer les petites pensions et encore moins celui l'emploi des seniors. Ce projet consiste à reculer l'âge de départ en retraite pour respecter cela vient d'être dit, la règle des 3% qui ne correspond plus à grand chose dans l'époque où nous sommes là même austérité qui a conduit les gouvernements successifs par exemple à ne pas remplacer des départs en retraite dans la fonction publique et qui a déséquilibré les finances des retraites justifie aujourd'hui de nouvelles régressions sociales. Cela fait près de 10 ans que la Commission européenne demande à la France de réformer le système de retraite et de reculer l'âge de départ. Aujourd'hui cette en contrepartie du plan de relance européen accorde qui a doté de 40 milliards. Pour la France que le gouvernement s'engage à réduire à la fois les droits à l'assurance chômage et à réformer notre système de retraite. Je rappelle que le projet de loi de finances pour 2023 à supprimer, entre autres, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui constituait une une ressource essentielle pour les collectivités territoriales, puisqu'elle a représenté en 2021 5,7 milliards d'euros pour le bloc communal et 3 8 pour les pour les départements d'ici à 2024 ce sont 16 milliards d'euros en moins pour les entreprises et l'État soit exactement le montant du déficit du système répressif, comme évoqué par le gouvernement. Je vous remercie. Oui c'est un avis défavorable, parce que c'est la loi organique qui défini la forme du tableau, vous ne pouvez pas rajouter une colonne comme cela. Merci. Si Monsieur le Ministre. Je vous remercie. Explications de vote Madame Cohen. merci madame la présidente. 2 ans de plus donc 2 ans de vie volée qui doivent permettre de réduire les dépenses de retraite pour te dire les engagements du gouvernement à respecter le totem du 3% du du 3% du déficit public, ce fameux 3% dont les économistes s'accordent à dire qu'il ne correspond à aucun indicateur économique sérieux. La règle du 3% qui justifie toutes les régressions sociales depuis 30 ans est né sur un coin de table, mes chers collègues récemment l'ancien haut fonctionnaire de la direction du budget qui en est à l'origine précise même un journaliste que ce chiffre de 3% n'a aucune réflexion théorique, alors pourquoi 3% lorsque 1000 ans en 1982, le président de la République de l'époque François Mitterrand rencontre des difficultés économiques avec un déficit qui atteint les 100 milliards de francs. Il a demandé à ses conseillers de trouver un chiffre en pourcentage, plus accessible. Après avoir hésité avec 2% c'est le chiffre de 3% pour le maximum du déficit public qui a été retenu. C'est ensuite un certain Laurent Fabius ministre de des finances qui a repris ce chiffre avant lui-même d'être pris dans le traité de Maastricht, devenant un des critères pour pouvoir intégrer la zone euro. Ainsi donc, parce qu'il y a 40 ans, le chiffre de 3% a été retenu et pas celui de 4%. Par exemple vous allez sacrifier 2 années de vie à nos concitoyennes et nos concitoyens votre réforme comptable de trompe personne ni les 9 organisations syndicales de salariés ni les 3 quarts des Français ni les 93% d'actifs qui s'oppose à votre coup de force et qui seront présents. Je peux encore vous le rappeler une nouvelle fois, si vous n'avez pas enregistré la date, le 7 mars. Merci madame Cohen Madame Lienemann. il fallait en trouver un. Hop oh mais comme je vous l'avez dit tout à l'heure, ça devait être valables jusqu'au passage de l'euro. Et ensuite. Rendons à François Mitterrand, ce qui est à François Mitterrand, il avait toujours expliqué que la deuxième étape devait être accompagné d'un gouvernement économique de la zone euro qui devait définir le cadre macroéconomique de manière pluriannuelle et c'est Jacques Chirac, son gouvernement qui a négocié le traité d'Amsterdam sans introduire l'arbitrage un gouvernement économique en reprenant pur sucre ce qui étaient des critères de convergence pour être des critères ad vitam eternam. Et ça pèse très lourd, parce que ça a été une façon une vision malthusienne du développement de l'Union européenne. Je rappelle que depuis cette période la croissance moyenne en Europe est la plus faible du continent du monde.

À ajouter un critère de la baisse des dépenses publiques. Excusez du peu. C'est exactement le débat qu'on a. C'est-à-dire est-ce qu'on dépense, on baisse la dépense publique ou est-ce qu'on trouve des recettes pour limiter le déficit public. Or la logique libérale de financiarisation de la commission a veillé à dire non seulement il faut que vous baissiez le déficit mais la dépense. Si bien qu'au sommet de Barcelone. Il a été écrit noir sur blanc qu'il fallait baisser la dépense publique que l'âge moyen des retraites dans l'Union européenne et ça c'était en 2002, l'âge moyen de départ en retraite dans l'Union européenne devait. Rapidement atteindre 63. et qu'il fallait développer les fonds de capitalisation, excusez du peu. L'Union européenne à matrice et une certaine vision que vous avez dit reprise et mais. On pénalise les Français. Merci. Madame Rossignol. Vous avez à la parole même la présidente. Je vais poursuivre ce que disait il y a un instant Marie-Noëlle Lienemann parce que des collègues pourraient penser que ce débat en fait est un peu périphérique au débat que nous avons sur. La défense de nos systèmes de retraite et le droit pour les salariés à une retraite suffisamment longue pour qu'ils puissent en profiter. Et le débat sur Maastricht la dette les critères et la baisse des dépenses publiques, or nous en sommes au coeur de ce débat là si nous avons eu les différentes réformes sur les retraites. Ce n'est pas parce que les déséquilibres démographiques le justifiait. C'est parce que la compte le la la conjonction de la baisse des dépenses publiques et des pressions sur le coût du travail et des salaires, nous ont conduit à réduire la masse salariale de ladite masse salariale réduisant les dépenses, les, les recettes de l'assurance vieillesse et le débat sur les déficits. Sur les les critères de Maastricht, c'est le débat que nous avons tous les jours, mes chers collègues, dans cet hémicycle un jour nous parlons de l'hôpital de de son état de la difficulté qu'ont les personnels de la difficulté qu'ont les médecins un jour nous parlons de la justice, de la difficulté qu'ont les justiciables à se voir avoir jugé leur leur litige de la difficulté des magistrats de l'engorgement des tribunaux. Un jour, nous parlons des transports du rail de la difficulté qu'ont nos concitoyens à prendre un train le matin quand ils espèrent pouvoir aller travailler avec tous ces débats-là, ce sont les débats qui sont la conséquences des choix qui ont été faits au moment la construction de l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un espace libérale destinée à faire baisser les prestations sociales et les services publics et nous sommes dans le débat sur les prestations sociales des services publics, donc nous voterons cet amendement. Merci cher collègue. Monsieur Savoldelli. Merci madame la présidente, monsieur Ministre mes, mes chers collègues. C'est c'est pas un débat de sémantique. C'est un débat politique. On a là, y compris toutes les interventions qui succède le montre et comme vous avez beaucoup parlé ou pas assez de la dette publique. C'est normal qu'on s'attarde sur les mots. La dette publique en 2021. Ah s'élevait, monsieur le ministre, à 2813 milliards au sens du traité de Maastricht. Soit 112 5 % du PIB. Ministre, la dette publique au sens de l'Insee. N'est plus que de 2522 milliards d'euros, soit 101,2 point de PIB. Et mieux encore en 2021 toujours, la dette publique nette au sens d'Eurostat et l'OCDE n'est plus que de 2174 milliards, soit 87% du PIB. Donc ce qui vient d'être débattu et ce qu'a expliqué la présidente Assassi c'est pas un tour de passe-passe des sénatrices et sénateurs communistes. C'est une autre méthode de calcul. C'est pour ça que les mots ont du sens. Madame la rapporteure et que c'est pas un amendement mineur et secondaire parce qu'il y a une autre méthode de calcul qui consiste simplement à déduire les actifs ou plus largement la valeur financière nette pour Eurostat et les engagements financiers nets pour l'OCDE, donc il y a une question de logique. C'est pas qu'une question comme ça de petits mots et de petits amendements. Parce que ça nous renvoie quand même à un niveau de la dette par rapport à notre PIB voyez à 3 calcul différents. Donc c'est pour ça qu'il faut voter cet amendement. Merci. Alors si il y a même souri à monsieur Reina. Monsieur le président vous avez la parole. Merci. Oui je voulais revenir, je trouve que ce débat sur Maastricht et tout à fait intéressant et sur la façon en fait de faire ses équilibres. C'est le point qui nous occupe aujourd'hui, mais pas qu'aujourd'hui ça a été rappelé par Laurence Rossignol, c'est vraiment un enjeu permanent sur quelques sujets récents finalement. À cette difficulté déjà de l'équilibre a donc rajouté. La, la volonté de, de baisser les impôts dans notre pays dans une période qui, sincèrement, ne s'y prêtait pas ça au moins on peut le reconnaître parce que avec des crises successives. Comme nous avons eu, est-ce bien le moment de baisser les impôts. Alors je ne reviendrai pas sur l'impôt sur Liès fait la démonstration a été faite entre 2006 et 2023 il y a donc une augmentation encore heureux. C'est même pas l'inflation, mais si on regarde bien les choses. Bon donc restons restons calme sur le sujet enfin. Je vous dirais sur ce point de liesse quand même et vous nous le savons tous, tous ceux qui ont dirigé une entreprise savent que c'est pas parce qu'on baisse l'impôt sur les sociétés. Que l'on a des profits qui augmentent, c'est pas la réalité. La baisse de l'impôt sur les sociétés permet éventuellement d'investir davantage a ensuite ayant plus investi, on peut avoir des bénéfices, donc ce n'est. C'est tout à fait sans lien, je voudrais dire que c'est la même chose pour la CVAE la. On enlevé 20 milliards personne est capable de nous dire où ils sont passés personne et je rappelle juste ici que le Parlement a voté contre à l'Assemblée nationale. Ils ne l'ont pas vu et. Au Sénat, nous avons voté contre et malgré tout la CVAE continuent à être supprimés. Et donc et c'est un problème parce qu'on pourrait effectivement là aussi récupérer facilement quelques milliards. C'est une évidence et personne ne nous a prouvé pour la première partie des 10.000 et 20 milliards correct et supprimer que ça avait eu quelque effet que ce soit enfin je termine avec le dernier point sur quand même le balancier pour les habitants. Vous avez d'un côté on a enlevé la taxe d'habitation qui n'étaient pas payés par 30% des moins aisés de notre pays et de l'autre côté hé bien maintenant on va sanctionner tout le monde mais vous des retraites. Merci monsieur le président je mets aux voix l'amendement 3793 qui a reçu 2 avis défavorables qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe communiste citoyen et républicain sur l'article liminaire. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56. Explications de vote.

qui dit tranquillement les dépenses de retraites ne dérape pas, elles sont relativement maîtrisée dans la plupart des hypothèses, elle diminue plutôt à terre mais dans l'hypothèse retenue par le gouvernement, elle diminue très très peu mais un peu à terme. Alors je vais aussi citer monsieur Brun qui s'est exprimé devant l'Assemblée nationale. En tout cas les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat et il explique qu'il ne devrait pas y avoir de sol négatif si les dépenses reste constante par rapport au PIB. C'est là où il va y avoir des évolutions qui ne sont pas intuitive et il explique ce déficit par 3 phénomènes clair dont les 2 principaux sont les suivants. Tout d'abord, la baisse des dépenses de retraites, de l'État employeur pour ces fonctionnaires alors que ces cotisations. Représentent 15% de l'ensemble des cotisations versées quand les fonctionnaires ne représentent que 8% de l'emploi total 2ème a un effet Cnracl, c'est son expression concrètement une baisse des rémunérations des fonctions publiques territoriale et hospitalière dans les rémunérations totales cette diminution serait causé tant par une baisse de rémunération qu'une baisse des effectifs. En résumé, le déficit et creuser car ceux qui cotisent le plus cotiseront moins en proportion de la somme des cotisations. Monsieur, vous pourriez au moins reconnaître que ce sont bien aussi les restrictions sur l'emploi public qui génère le déficit annoncé du système de retraite et vous pourriez aussi reconnaître que vous projetez. Des économies non seulement sur les retraites en allongeant l'âge de départ mais également sur toutes les administrations publiques par la diminution du nombre de fonctionnaires d'État hospitaliers et territoriaux, hospitaliers territoriaux car à terme ce sont eux, c'est dans l'article liminaire qui contribueront le plus à la diminution des déficits publics. Merci cher collègue. qui ont soulevé un certain nombre de questions, on a même eu des réponses du ministre-sur d'autres amendements qu'on étudiera plus tard. Qui n'avait rien à voir avec la discussion en cours mais on avait eu, on a quand même une absence de réponse sur une, sur un certain nombre de choses notamment sur la sincérité du véhicule législatif qu'on est on qu'on utilise. On va rappeler les la la chronologie, le 29 novembre ici ont voté un PLFSS. À peine un mois plus tard, le 10 janvier, ont présenté une réforme qui concernait ce Plfss mais donc on doit le rectifier dans l'urgence parce que ça facilite le gouvernement pour nous corseter le débat et puis là on vient d'apprendre que vous dites à l'Assemblée nationale, c'est mon collègue Savoldelli qui l'a dit. Le là on on se base sur le texte de la loi de programmation de la des finances publiques votée au Sénat. Vous dites ça à l'Assemblée nationale et vous nous dites-nous ici non non ce sera le texte initial que qui n'a pas été voté à l'Assemblée. Donc on est sur quelque chose d'assez floue d'assez insincère, on n'a pas eu de réponse sur la trajectoire d'embauches dans la fonction publique qui a été soulevée par exemple de mes collègues. Même mon collègue sénateur du Rhône n'a pas eu de réponse sur l'avenir le la capitalisation on a, on ne sait pas si c'est le projet futur du gouvernement comme ça a été soulevée par son de mes collègues aussi et puis on a toujours pas la réponse de mon collègue jeune sénateur. Breuiller sur la note du Conseil d'État qui vous refusez de rendre. Donc on est encore un peu sur notre faim, dans le début de ces débats, je vous remercie. Madame Poncet Monge. Les 3,1 milliards des mesures sociales qui sont un mensonge. Et ramener donc vos mesures à 3 milliards sur 18 milliards. Donc vous avez dit que nous étions nous nous basons sur la loi de programmation des finances publiques ce texte qui prévoit dans ses articles 17 avant de cantonner les dépenses des branches de la Sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse à 21,8% du PIB de 2023. Juste ce dans sa version du Sénat. Ça a été dit la loi de programmation prévoyait un objectif de réduction globale des effectifs de la peur, fonction publique de 5% soit 120.000 postes. Cette réduction et c'est pour l'avenir. Nos discussions. Futures est en concordance avec la Convention EPR que vous favorisez sur lesquelles vous vous basez qui que sur lequel s'appuie le gouvernement qui prévoit un désengagement de l'État grevant les recettes de la Sécurité sociale et justifiant la réforme injuste dont on va discuter cette convention l'EPR. c'est pas une bonne. C'est pas c'est pas une bonne convention s'appuie sur une baisse de la rémunération des fonctionnaires, ça a été dit de 11% et une baisse des recrutements. Alors que si aucun décrochage organisé déficit serait réduit de 3 milliards. En conséquence, donc nous ne voterons pas cet ce, cet article préliminaire et les Français doivent savoir que la réforme des retraites dont parle ici rejoint une politique globale d'austérité qui va aggraver l'offrent des services publics, ils doivent savoir l'ampleur et la teneur de ce projet délétère sur l'ensemble des administrations publiques. Merci, cher collègue, la parole est à madame ah pour s'opposer. Merci madame la présidente. Henri Sterdyniak, membres des économistes atterrés. Dans une note présentée préalablement aux annonces du gouvernement, explique l'importance de la politique d'emplois publics pour le financement des retraites. Le corps reprend les hypothèses fournis par la direction du budget, le nombre de fonctionnaires sur fixe sauf les 15.000 emplois dans les hôpitaux. Promis au Grenelle de la santé, la nécessité d'embauches dans l'éducation, la santé, les soins aux jeunes enfants et aux personnes âgées dépendantes, la culture sont oubliés. De 2022 à 2037, l'indice de la fonction publique perdrait 8,3% au pouvoir d'achat, alors que le pouvoir d'achat dans le privé augmenterait lui de 12,7%. Aucune leçon n'est tiré de la dégradation de l'attractivité des emplois publics. Compte tenu de ces de ces hypothèses, la part du traitement des fonctionnaires dans la masse totale des rémunérations passerait de 15 en 2022 à 7,8 en 2037. Merci madame la présidente. Explications de vote effectivement sur cet article liminaire. Rappelé que contre l'avis des organisations syndicales et malgré l'opposition des Français qui se mobiliseront encore massivement mardi prochain dans tous les territoires et ce ne sera pas la fin du monde. Le gouvernement s'obstine à vouloir reculer l'âge légal de la retraite à 64 ans. Nous nous opposons. À cette réforme injuste qui n'est pas utile en l'état et brutal qui va pénaliser en priorité les femmes et tous ceux qui ont commencé à travailler tôt cette réforme. Brutale car elle va s'appliquer immédiatement, dès 2023, la retraite c'est une nouvelle vie, elle se prépare s'anticipe pour faire place à des projets personnels familiaux. Eh bien non. Ces Français qui devait partir à la retraite cette année, nous ne pourrons pas. Puisque nous sommes ici pour débattre et surtout pour dire la vérité aux Français, il faut avoir le courage de l'avouer. En réalité, cette réforme va créer encore plus de précarité et de pauvreté. Et aussi sur cette réforme, nous avons tout entendu le président comme la Première ministre nous au moins m'expliquait qu'elle permettrait de dégager des marges de manoeuvre pour financer d'autres politiques publiques, on en a parlé depuis quelques heures maintenant parce que c'est essentiel de dire aux Français ce qui on est véritablement de cette réforme, ce qui nous ont dit ce que vous vous nous avez dit démontre bien que le problème n'est pas les retraites, mais les finances car là encore, comment expliquer que ces économies sur le dos des travailleurs changent les paramètres de nos finances publiques. Quand on parle d'économiser 10 à 15 milliards par an. Tout ceci n'est pas sérieux et encore moins de parler de faillite à l'image du ministre Atal. Les Français ne sont pas dupes lorsqu'ils entendent parler de déficits abyssaux pour faire croire que ces restrictions s'imposerait pour sauver le système. La réalité c'est plutôt que certains déficits sont parfois volontairement entretenu. Il en est ainsi de la non-compensation des allégements de cotisations décidée par l'État pour la sécurité sociale. Ainsi, au travers de ses arguments, je dirais, nous pourrions en discuter plus longuement. Les raisons. Sont toutes claires pour expliquer que nous voterons contre 7h. Cher Merci madame la présidente, messieurs les ministres. Vous aurez compris que le groupe socialiste, écologiste et républicain votera donc contre cet article liminaire. et peut être que ça convaincra certains qui avaient déposé un amendement de suppression qu'ils n'ont pas voté. J'ai pas bien compris mais. Ça regarde la majorité sénatoriale. En tant que telle. Simplement vous dire que pour nous ce sera le premier acte officiel pour refuser cette réforme impopulaire. Je crois que tout le monde peut en convenir.

parce que nous ne sommes toujours pas persuadé que c'est par cette méthode qu'on pourra équilibrer le système des retraites par répartition. J'en profite d'ailleurs pour. Rappeler que. En 2021, ce régime tant décrié a dégagé un excédent de 900 millions d'euros. Et qu'en 2022, il a dégagé un excédent de 2 milliards d'euros, certes. Je regarde les courbes comme vous toutes et vous tous et je sais que ça va pas durer mais il peut y avoir des bonnes années. C'est le cas, alors dans quel contexte sommes nous. Mes chers collègues. Aujourd'hui viennent de tomber les résultats. Du de grandes entreprises françaises CGM. CMA. 25 milliards d'euros. De bénéfices, 25 milliards d'euros, plus que les 19 ou 20 milliards d'euros de Total. Et vous vous obstinez à droite. Et à la droite. Il s'y présente élyséenne vous obstiner à ne pas vouloir faire contribuer qui auraient les moyens de contribuer pour équilibrer globalement les dépenses publiques dans notre pays. Eh bien donc nous voterons contre certains pratique liminaire comme le signe de notre détermination pour voter contre, globalement, cette réforme des retraites. Merci monsieur le président. La parole est à monsieur le Leconte. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues de de de ce débat et en particulier des, des interventions du ministre des Comptes publics tout à l'heure, nous avons bien compris. L'objectif de cette réforme. Faire des économies. Financer les baisses d'impôts qui ont été. Alignées été. Alignées les unes avec les autres depuis quelques années, financer les exonérations ou. Les allégements de cotisations sociales qui ont été mises en place progressivement et en particulier lors de la loi sur le pouvoir d'achat à l'été dernier. Alors voilà pour faire des économies. Hé bien c'est. 900.000 personnes. Qui doivent c'est une génération. C'est une année de départ en retraite, c'est à peu près 900.000 personnes. Hé ben c'est 900.000 personnes à qui on va dire ben désolé ce sera l'année d'après. évidemment comme ça on fait beaucoup d'économies on fait beaucoup d'économie parce que on Report on on reporte. Des pensions à payer et en plus comme on pose des conditions complémentaires les pensions seront plus faibles donc on fait doublement des économies sur le moment et après voilà c'est la seule motivation que vous avez. Et je voudrais dire à ce stade qui a d'abord une conviction. On l'a vu auparavant sur l'assurance. Sur l'assurance chômage. Si on veut maintenir un bon niveau de protection sociale. sociale. D'abord être l'affaire des partenaires sociaux et pas celui de l'État dont on voit ce qu'il fait avec la protection sociale, un outil pour mettre la main dessus et financer ses déficits, et ça n'est pas acceptable et la conviction que j'ai aussi quant au regard de l'évolution. De ce que représente les pensions dans le PIB en France, c'est-à-dire que ça ne va pas augmenter. Contrairement à ce que vous dites ça ne va pas augmenter et ça c'est une préoccupation parce que compte tenu de l'évolution de la population. Si ça ne n'augmentent pas. Ça veut dire qu'on va revenir à une situation qu'on a connu il y a 50 ou 60 ans que progressivement les personnes de plus de 60 ans redeviendront des personnes pauvres

Merci madame la présidente. La raison pour laquelle nous ne voterons pas cet article. A été. Déployé. Le régime des retraites n'est pas en péril. Le président du corps l'a souligné à de multiples reprises les dépenses de retraites sont stables depuis 2010. intérieur brut et toutes les études garantissent cette maîtrise jusqu'en 2070. Nous avons même cette année et pendant 2 ans. Des excédents. Qui. Montre qu'effectivement la situation est loin d'être catastrophique, nous avons. Un problème ponctuel, c'est celui du papy-boom du baby-boom. Il faut l'absorber. C'est en passe d'être fait, nous en sortirons assez rapidement et le régime retrouvera son rythme de croisière. Si le corps anticipe dans son scénario. Ce déficit entre 2022 et 2032, il sera entre 0 5 et 0 8 point du PIB. Ceci peut paraître important en valeur absolue mais faible en valeur relative. Une des raisons. Qui. Justifient les difficultés que nous rencontrons. Ce n'est pas une raison démographique c'est une raison politique c'est celle de la volonté d'appliquer à l'ensemble de la fonction publique. Une politique d'austérité depuis 2017. Cette politique d'austérité elle ce couple par ailleurs à un démantèlement progressif de la fonction publique en obligeant l'ensemble des administrations publiques de l'État, la fonction publique hospitalière, la fonction publique territoriale de recourir de plus en plus fréquemment aux contractuels. Or c'est ce qui déséquilibre aujourd'hui les possibilités. D'abondement. Les systèmes de retraite. C'est ce qui explique aujourd'hui aussi les difficultés de la Cnracl et quand on ajoute à cela

Chers collègues. Beaucoup d'arguments plaident déjà pour refuser cet article liminaire. Mais il faut bien regarder dans, comment se déroulent ces successions de réforme. Chaque fois le même scénario. D'abord on gonfle les déficits. On assèche les retraites les les retraites on assèche les recettes. Conclusion, le niveau des retraites et l'accès à ces retraites se dégrade. Et là arrive les publicités sur. Dont vous n'aurez plus de retraite alors ça donc prenez des assurances et le club en l'occurrence des fonds de pension. Et là, chers collègues de l'air, mais au moins vous avez l'avantage de vous dévoiler. C'est comme d'habitude. C'est le prétexte de sauver le régime des retraites. La réalité c'est que vous voulez des retraites minimales et une grande part de capitalisation tout cas croissante. Je voudrais insister sur le fait que, par ailleurs vos calculs financiers sont inexacts. Outre le fait que vous séché et que vous décidez pour des lustres que la contribution de l'État ne va pas, ça ne va pas augmenter au nom de quoi, vous pouvez décider aujourd'hui qu'on ne va pas augmenter le nombre de fonctionnaires jusqu'en 2037 au nom de quoi. Tout ça est très aléatoire mais surtout. Mais surtout. Vous n'avez et là je vous interroge Monsieur le Ministre. Combien évaluez-vous. Le nombre de seniors. Supplémentaires qui vont être dans la zone grise ni emploi. Ni retraite. Combien y aura-t-il de RSA. Combien y aura-t-il d'ASS. Combien y aura-t-il de seniors supplémentaires au chômage. À ma connaissance, les administrations ont évalué chaque année à 40.000 supplémentaires dans chacune de ces catégories. Si Madame Lienemann. La parole est au président Laurent. Merci madame la présidente. Je voudrais m'adresser à mes collègues LR avant tout passions vote sur une guerre parce que vous êtes très nombreux, mais visiblement condamnée au silence par un coup de baguette magique du président Retailleau j'imagine qu'il vous a demandé de ne rien dire survient. Alors je voudrais vous interpeller parce que après avoir entendu le ministre Atal. On a compris que sur le Haut conseil des finances publiques, c'est du bricolage intégral, on ne sait même pas ce que vous avez voté si c'est utilisé ou pas respecté ou pas. À propos des règles européennes. On sait qu'on va devoir les changer qu'elle n'existe pas mais on continue de les utiliser à tort et à travers un de vos collègues tout à l'heure Étienne Blanc a expliqué que l'article liminaire c'était n'importe quoi et que d'ailleurs il ne serait pas respecté à la, à l'arrivée il n'a d'ailleurs pas voter son propre amendement mais ça, ça le regarde. Mais. Tout ça ne vous ressemble pas jusqu'à quand vous allez voter ce grand n'importe quoi budgétaire. C'est quand même pas brillant pour des des grands spécialistes de la rigueur budgétaire. Vous allez continuer à ne rien dire. Alors nous ne sommes pas d'accord sur le fond, c'est clair. Vous voulez à tout prix. Arrivé au vote pour les 64 au parce qu'il y a cinq il y a que ça qui compte pour vous. Mais jusqu'à quand vous allez cautionner et la la méthode du gouvernement le 47 ans et tout ce qui va avec. Les calculs fabriqué de toutes pièces du gouvernement pour justifier statistiquement son projet de réforme. Est-ce que vous allez on a un mot, je vous pose la question. Continuer à laisser abaisser le Sénat de cette manière. Merci madame la présidente, messieurs les ministres. Cet article liminaire est essentiel au fond il monte que cette réforme n'a qu'un objectif, faire baisser les dépenses publiques pour respecter les objectifs du pacte de stabilité et de croissance mais il n'est pas admissible que cela se fasse au détriment de la santé et de la qualité de vie des Français. À un moment de sa vie, il est bon de pouvoir penser que l'on arrête le labeur pour vivre un autre rythme et 2 ans de plus à travailler, ce n'est pas rien, surtout pour ceux qui sont les plus abîmés par le travail. Mais ces décisions ont auront aussi d'autres conséquences. Ces jeunes retraités. Ce sont eux qui font la richesse de nos engagements associatifs. Ce sont souvent eux qui sont les conseillers municipaux qui nous élisent chers collègues ce sont eux aussi qui s'occupe des petits enfants quand hélas les places en crèche manque qui s'intéressent à la santé de leurs parents en grand âge parce que là encore le le manque de structures publiques et cruel et donc tous ces éléments-là ne figure pas dans le tableau de cet article liminaire ils auront pourtant des coûts sociaux et des coûts dans la cohésion sociale très lourd enfin je voudrais redire Monsieur le Ministre pourquoi ne publiez-vous pas ce texte. L'avis du Conseil d'État qui n'est pas un avis mais tu mets une note de synthèse et qui permettrait qu'ici nous sachions tous. Ce que vous savez tous parfaitement chers collègues à savoir qu'on utilise un véhicule législatif qui va empêcher et corsetée un travail hein. Une réflexion et un débat sincère sur les enjeux du travail car oui derrière la question des retraites, il y a d'abord les enjeux du travail et c'est d'abord de sacs nous devrions parler lorsque nous abordons ce débat donc Monsieur le Ministre, je le redis, les parlementaires ont droit à une information autre que la lecture des journaux. La parole est à madame le oui. J'ai également un doute sur la sincérité budgétaire ne cet article, il fait état d'une hausse de 400 millions d'euros de la branche. La branche vieillesse correspondant à des mesures d'accompagnement liées à la présente loi, notamment relatifs à la pénibilité toutefois pas de baisse de dépenses observé ni de hausse de recettes générées par les mesures de cette réforme, censée entrer en vigueur à partir de septembre au cours du précédent quinquennat. Le budget de l'État a été imputé à hauteur de 50 milliards d'euros par an suite à des baisses d'impôts au profit des plus riches et des grandes entreprises. Suppression de l'ISF, création de la flat tax et maintenant la fin de la CVAE. Le déficit prévu pour 2023 n'est pas la résistance la résultante d'un déséquilibre démographique mais un choix politique. Le conseil d'orientation des retraites prévoit un retour à l'équilibre à horizon 2050, avec un effort de l'État constant dans le financement des retraites à hauteur de 2% du PIB. Alors qu'Emmanuel Macron lui-même balayé la prétendue urgence financière dans son programme de 2017. Le sauvetage du régime redevient la justification central de la réforme pourtant la santé financière du système de retraite ne justifie aucunement le recul de l'âge légal le départ à la retraite et l'augmentation de la durée des cotisations qui aurait des conséquences sociales désastreuses, les projections du gouvernement repose sur la convention dite équilibres permanent des régimes qui suppose une diminution progressive de l'effort de l'État dans le financement du système de retraites découlant de la baisse de l'emploi public dans l'emploi local comme les employeurs publics ont des taux de cotisation supérieure au régime général du privé. Moins il y a de fonctionnaires, moins l'État participe au financement du système de retraite et plus on équilibre menacée par ce vote contre contre cet article. Préliminaire nous manifestons donc notre position générale au projet de réforme des retraites. Merci, cher collègue, la parole est au président rénale. Moi je voudrais dire à ce soir quand même. Que on est au début d'une phase d'étude de ce texte. Mais après une période tout à fait particulière. Ça fait 6 ans déjà 6 ans. Qu'on nous parle de réforme des retraites, une paille. Je voudrais pas qu'on oublie quand même que chaque fois, nous avons affaire à une réforme géniale chaque fois.

ça imploser en trois mois. Juste en réfléchissant un peu, en montrant que certaines professions été totalement oubliée. Juste les enseignants par exemple il y a juste quelques millions d'enseignants, une paille. Bon et donc tout d'un coup ça capote c'était génial ça a capoté. Ensuite, on nous dit 2ème mandat, on nous dit oui, retraite à 65 ans, retraite de type paramétrique bon lance ça. Et on commence à à démarrer l'opération. Très bien. Et puis on sent que ça prend pas et s'en prend pas parce que il faut une majorité juste une paille. Il faut une majorité pour la voter et finalement conclu par quoi non plus par un projet du gouvernement mais finalement par le projet de la majorité sénatoriale, c'est quand même très particulier. Un gouvernement qui fait ça d'ailleurs je voudrais dire gobant toutes l'autre jour de la de la DG. Moi je me suis étonné que le président Retailleau ne parle pas

Je le regrette et puis ensuite quand même on est passé de Bruno Le Maire qui disait la vérité c'est budgétaire, bon on l'a fait taire. On l'a dit non non c'est pour le bien des retraités.

parce que quand même si j'ai bien compris, vous me dites si je me trompe article liminaire, c'est l'état des prévisions. C'est l'état du sol structurelle et l'état de la prévision, donc c'est sérieux quoi, comme dit le ministre est crucial. Alors moi je vais vous dire c'est que là on est dans une logique alors soit la partage. Totalement et on y va. C'est-à-dire on fait comme pour l'assurance chômage. Version apocalyptique du gouvernement. On fait une réforme avec un excédent de 4,1 milliards mais c'est catastrophique. Et on fait perte des droits. Aux travailleurs et là c'est la même chose. Et là moi je m'adresse à mes collègues de droite vous nous répétez à chaque fois à chaque projet de loi de finances, vous les communistes. L'entreprise vous y connaissez rien, vous défendez par l'entreprise. Hé ben moi je vous lance un défi, je vous lance un défi, je vous lance un défi fait pareil avec la dette publique faites comme dans les entreprises privées, c'est très simple, je vous donne la méthode vous avez soustraire les actifs, vous connaissez l'entreprise moi aussi je la connais, vous soustrayez les actif et le passif. Et qu'est-ce que ça s'appelle dans le langage dans un Chapatte d'un patron, ça s'appelle le bilan de l'entreprise. Et ben donc c'est très important. L'article liminaire parce que la dette publique de la France c'est pas 112 5 % de PIB, c'est 87% de PIB. Et là on a un problème on peut avoir un avis différent sur plein de sujets mais on ne peut pas accepter qu'on nous vend des mensonges et des comptabilités qui sont pas juste voilà c'est ça le problème parce que derrière c'est l'économie. Allez voir les fonctionnaires, vous croyez que je vais faire comment. Dans mon département et dans le vote quand il manque des enseignants. Ils sont où là dans nos débats et les contractuels dans la fonction publique, il y en a plus de 600.000. Vous savez ce que c'est leur vie 41% sont CDD, 68% des contrats de moins d'un an dans ce qu'ils versent à leur régime il y a 25% des contractuels de la fonction publique si ne va pas l'Ircantec. Ils n'ont pas de retraite complète. la parole est à monsieur Redon ça reste. Alors le prévisions on parle hypothèse et donc pour revenir donc sur les hypothèses que l'on peut retenir. On peut choisir peut-être les hypothèses les plus crédibles. Parmi les hypothèses de croissance économique la plus crédible c'est celle qui est à plus 1,3%. Elle est cohérente cohérente avec des projections de courts termes du gouvernement ainsi qu'avec les estimations de long terme des différentes institutions internationales, en ce qui concerne le taux de chômage retenir une hypothèse de 7%, à long terme est un choix prudent et réaliste. En ce qui concerne la participation de l'État au système de retraite. Il s'agit d'un choix avant tout politiques, il peut décider de réduire ou de maintenir son niveau de dépenses en faveur des retraites votre gouvernement retient d'autres hypothèses économiques il choisi unilatéralement de réduire sa participation au système de retraite, hypothèse qui aggrave un Campus. Le déficit du système ce choix politique ne signifie pas signifie une baisse des rémunérations réelles compte tenu de l'inflation. Un ralentissement voire un gel des pensions des fonctionnaires un recul de la participation de l'État implique aussi moins de financement des mécanismes de solidarité et de retraite et des systèmes de retraite et donc en ce qui concerne le besoin de financement pour en avoir une juste appréciation. Il faut regarder donc à court terme mais à moyen terme et aussi une tendance à long terme. Ainsi, si l'on considère à la fois un taux de croissance de 1,3%, je le disais, un taux de chômage de 7%. On peut dire, alors que le besoin de financement s'en 2027. 7 milliards d'euros si l'État maintient sa participation. 9 milliards d'euros si l'État réduit sa participation en 2044 milliards d'euros si l'État maintient sa participation 18 milliards d'euros si l'État la réduit et à long terme entre une stagnation sans dérive du besoin de financement. Si l'État réduit sa participation et une amélioration, suivi de l'excédent de financement. Si l'État maintient sa participation. Dit autrement, le besoin de financement du système de retraites évolue au sein de l'intervalle qui dépend directement des choix politiques. Que fera l'État. Pour toutes ces raisons et elles sont nombreuses, nous voterons effectivement la suppression de cet article. Pardonnez-moi. Les collègues ont tous donné les raisons. Fort. Va mais légitime pour. Voter contre cet article liminaire, j'ai une autre raison en m'adressant. À mes collègues de la majorité sénatoriale. Après 6 ans de présence ici. Je croyais qu'il y avait quelque orgueil voir quelle fierté d'appartenir à cette maison là pour de sombres calculs qui sont les vôtres vous avez décidé d'accompagner le gouvernement en piétinant les lois du Parlement. Vous avez l'impression que, en faisant cet abus de majorité. J'allais presque dire une majorité sénatoriale tyrannique contre la minorité que nous sommes, vous servez vos intérêts. Mais oui alors que vous aviez la possibilité de 20. Gouvernement qui quémande. Votre accompagnement de faire plier le gouvernement et je crois comprendre que vous pourriez avoir une forme de conservatisme éclairé. Je ne comprends pas cet abaissement et cette faiblesse. Parce que vous voulez, vous n'êtes pas au gouvernement, vous pensez que ce sera la retraite Retailleau. Franchement je trouve ça un peu étonnant après 16 ans de présence. La raison pour laquelle je demande un sursaut de lucidité, pardonnez-moi, ça se fait que vous aurez pas blessé de dignité sénatoriale. Merci la parole est à monsieur, si. Merci cher collègue. Il se trouve que je suis un, je fais part parmi les les anciens dans cette honorable assemblée. Et très honnêtement, c'est bien la première fois en plus de 20 ans. Que je vois un débat de cette qualité. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte. Que nous sommes, nous À cette heure-ci. De donner la même impression que le peuple français retient de l'Assemblée nationaux. Ainsi. Ah. À ceci près. Non attendez, attendez, à ceci près, j'ai entendu un journaliste tout à l'heure dans la salle des conférences. Faire ses observations et nous dire que finalement, ici au Sénat, c'était l'obstruction cordial. Je trouve que le mot était bien choisi. Mais est-ce que vous vous rendez compte quand même que de défendre 60 ou 80 amendements identiques de les défendre tous les uns après les autres, mais quelle idée, cela donne. Aux Français qui sont très soucieux de cette question des retraites. Il y a un véritable problème. Alors. Je ne sais pas ce que vous cherchez, enfin je le devine, c'est finalement de faire en sorte que nous n'arrivions pas à la fin du débat et au vote de cette loi peut être. Mais. De mon point de vue, je vous le dis très tranquillement, mais tout cela ne rehausse pas l'idée que les les Français peuvent se faire du Sénat. Alors. J'ai, j'espère, j'espère que vous allez vous ressaisir, merci. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Marie.

et pour tout vous dire nous dépôt nous défendrons tous nos amendements. C'est notre droit le plus strict entre parlementaires. Nous n'avons pas à recevoir de leçons de qui que ce soit par rapport à ça et nous le ferons d'autant plus que depuis des semaines. des milliers et des milliers de Français manifestent. Dans avec une dignité remarquable. Vous ne les entendait pas, donc nous, nous allons être la chambre d'écho des Français et des Françaises qui manifestent depuis plusieurs semaines et que vous ne souhaitez pas écouter et à travers ces amendements, c'est ça que nous défendons et que nous continuerons à défendre parce que cette réforme allait profondément injuste. Allez profondément brutal et c'est normal que nous soyons là au combat avec tous les bancs de la gauche pour défendre justement le peuple français qui souffrent qui va souffrir à cause de ça. Cette réforme si elle est adoptée et c'est l'honneur du Parlement justement de pouvoir défendre ça dans l'hémicycle dans un, dans un délai contraint que vous acceptez vous-même que vous acceptez, qui est imposé par ce gouvernement et vous auriez honneur justement à intervenir dans ce débat nous avons attendu une seule prise de parole mais intervenait c'est votre réforme défendait la justifier la. Argumenter, c'est ça le Parlement c'est pas de se taire. C'est pas d'avoir un bas le bâillon Retailleau sur la bouche, c'est de pouvoir intervenir défendre vos arguments fait comme monsieur Pradié

La parole est à Madame Rossignol. d'avoir d'abord d'avoir eu l'audace de prendre la parole. Puisque, en effet c'est le la première fois quasiment que nous avons entendu et je voudrais lui dire assez clairement que effectivement vous avez raison. Quelle image on les Français du Parlement mais aussi du gouvernement et globalement de ceux qui gouvernent ce pays de dirige le représente alors que depuis des semaines. Ils disent par tous les moyens possibles, mais par des moyens pacifiques légaux. Il s'exprime dans des manifestations qui sont des manifestations aussi massive que sereine. Il ne s'exprime dans les enquêtes d'opinion. Il s'exprime par des mouvements de grève des mouvements sociaux, ils disent nous sommes 67 Français sur 10 ne veulent pas de cette réforme. 7 Français sur 10 ne veulent pas cette injustice. Alors après il y a 2 options dans les dans l'exercice démocratique soit l'option qui a fait qu'a choisie le gouvernement qui consiste à dire on vous entend pas ou mieux vous avez rien compris, on va vous expliquer d'ailleurs plus explique-moi les gens comprennent ou plutôt plus ils comprennent que ce qu'on leur a expliqué, n'était pas la vérité. Et puis il y a l'autre option qui consiste à dire nous allons traduire au Parlement ce mouvement pacifique de la population et, voyez-vous. Vous ne nous dites tout comme d'hab beaucoup d'amendements. Oui c'est vrai mais vous savez la concession de 58 donne une armurerie exceptionnel oh majorité gouvernementale et parlementaire au gouvernement et à la majorité sénatoriale pour tordre le bras des des oppositions. Et de la majorité des Français, voire même je me demande si à l'Assemblée nationale. Ils ont pas eu un problème de majorité à l'Assemblée nationale pour recourir à la méthode qu'ils ont choisi. Et nous, opposition. Nous avons quelques moyens, nos convictions, notre parole notre droit d'amendement et nous on useront jusqu'au bout.

j'écoute ce débat et je pense qu'au contraire, je pense que le Sénat, je pense que le Parlement ce soir il sort particulièrement grandi parce que oui il y a eu toute une liste d'amendements effectivement qui pouvait se ressembler. L'ensemble des arguments qui ont été donnés par tout le monde. Avait une vraie argumentation mais en face, moi j'ai rien entendu des ministres qui sont restés muets. Les seules réponses qu'on a pu avoir ses sur des amendements qui sont Georges qui vont arriver sur lequel on a même pas encore pu on a quand même pu débattre. On a demandé des éléments, on les a toujours pas on nous renvoie pareil. Ah je ne sais quand. Et puis de votre côté, cette réforme que vous voulez construire cette réforme que vous souhaitez de vos voeux, qui est, j'ai l'impression, votre seul projet votre seul projet de faire travailler les gens plus étroit les C'est ça le Parlement c'est ça c'est qu'on débatte, c'est qu'on comprenne vos arguments, c'est qu'on comprenne aussi justement je pense les erreurs que vous pouvez faire. Alors que là voilà on a un Parlement à plat qui ne débat pas. Et puis derrière ça il y a aussi ce fantasme de l'Assemblée nationale, on l'a eu hier soir avec les ministres ont tenté, essayer de faire attention. Voilà, essayer de faire monter un petit peu la la sauce et puis là vous êtes un petit peu déçu en fait vous êtes un petit peu déçu par la qualité des débats qu'on peut avoir par les arguments qu'on peut avoir. Alors moi j'attends de votre part d'avoir la même qualité de débat. Je vous attends. Prenez la parole. Expliquez-nous votre projet et là oui on aura du vrai débat et la oui le Sénat sera mis en avant. Merci. Si Monsieur le Président. Madame de La Gontrie. Vous avez la parole. Merci madame la présidente. Si pour un rappel au règlement, se fonder sur l'Arctique 46 bis du règlement. J'ai écouté Monsieur. Je suis stupéfaite. Parce que. Ce débat est important. Et. Vous évoquez le fait que les Français auraient si le suivait l'image. D'un débat qui serait d'aussi mauvaise qualité je le comprends. Dans votre bouche que celui de l'Assemblée nationale. Et je pense que si c'est le cas. C'est de votre fait. Parce que nous sommes dans une situation où la majorité de cette assemblée ne participe pas au débat. Et totalement passive discute. On ne sait pas très bien pourquoi vous êtes là puisque de toute façon monsieur Retailleau vote pour l'ensemble de son groupe au point que tout à l'heure, certains auteurs d'amendements de suppression de l'article n'ont même pas pu le voter. Donc je pense que c'est à vous de vous ressaisir de participer au débat de dire pourquoi par exemple vous vouliez maintenir l'article liminaire pourquoi par exemple vous souhaitiez laisser les termes de Maastricht et pourquoi depuis le début vous souhaitez défendent ce texte donc nous retiendrons et nous le diront et nous le répéterons à l'extérieur qu'ici dans cette chambre. La droite, majorité du Sénat n'a jamais participé à ce débat et a donc été totalement passive. Chers collègues. Donner de ce rappel au règlement. La parole est à monsieur Fabien Gay. Merci madame la présidente pour une explication de vote. Merci madame la présidente. Messieurs les ministres, mes chers collègues. Bon. Avec mes enfants à la maison je joue au roi du silence. À la maison, ça fait du bien. Mais dans l'hémicycle. C'est moins bien. Et je le dis avec une pointe d'humour mais. Faut qu'on fasse extrêmement attention les uns et les autres. Il faut. François. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais revenons à l'essentiel, je pense qu'il faut faire extrêmement attention. Il ne faut pas scier la branche sur laquelle nous sommes assise. J'ai écouté assez attentivement hier. Chaque oratrices et orateurs. Sur. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale sur la une caricature de devrait s'organiser les débats. D'abord le droit d'amendement et constitutionnelle. Et ici, nous sommes là pour parler et pour faire la loi et pour la fabriquer. Il faut une confrontation d'idées et nous vous le disons chacun avait nos mots mais nous sommes prêts au débat assez argumenté mais il faut que, en face. Aussi. Il y a une réaction sinon on va passer 12 jours oui, extrêmement difficile pour les uns comme pour les autres mais attention aussi. Si vous continuez à dire attention pas d'obstruction et cetera viendra une réforme constitutionnelle. Moi je suis arrivé il y a pas si longtemps que ça. On avait déjà deux minutes 30. Aujourd'hui c'est plus de que deux minutes et en faisant ce que vous êtes en train de faire, vous allez ouvrir la porte en réalité à réduire le droit d'amendement et c'est-à-dire si nous en venons sur une réforme du Parlement. C'est en réalité nous mettent de plus en plus en difficulté et ensuite ça sera réduire le nombre de parlementaires et cetera et cetera donc si on pas la broche agissons débattons et argumenter puisque vous avez beaucoup d'arguments pour la retraite à 64 ans. Nous vous entendons. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Vallée. Merci madame la présidente, je voulais saisir l'occasion de l'intervention de notre collègue Bruno Sido pour revenir sur. Un état d'esprit sur un vote qu'on a eu il y a quelques semaines et au cours duquel je pouvais parfaitement comprendre ces arguments là nous avons des collègues qui nous ont expliqué. De l'autre côté de l'hémicycle, qu'il n'y avait pas d'un côté ceux qui pouvaient être fiers de leur vote et ce qui devrait, par définition, avoir honte de leur vote. Hé bien de la même façon. Nous sommes dans une assemblée où on pratique j'espère une forme de confraternité je dis aussi à l'attention du gouvernement. Il n'y a pas là des gens bien élevés. D'un côté et des gens qui ne se comporterait pas correctement ou à qui on ferait par avance le procès d'intention de ne pas de bien se comporter dans un débat l'obstruction par silence ou l'obstruction mutique est aussi une forme d'obstruction et c'est une forme d'obstruction qui nous empêche d'entende les arguments des uns et des autres. Parce que moi ce qui m'intéresse c'est pas de nous prendre par avance des leçons de maintien. Ce qui m'intéresse et n'entendent, Bruno Retailleau et pas d'avoir l'impression n'entendent Nadine de Rothschild. Nous sommes des gens polis bien élevés, mon collègue. Du département de la Charente-Maritime qui siègent dans votre groupe et qui me connaît bien, c'est que je ne me mouche pas dans la nappe. Quand vous croisez la présidente Assassi au restaurant du Sénat. Elle n'a pas le couteau entre les dents. Et donc, je vous suggère toute de suite, d'éviter d'être sur ce registre-là parce que vous viendrez d'autant plus vite sur les arguments de fond et surtout je le dis dans l'intérêt de notre haute assemblée. Et pour que l'image que nous souhaitons tous donné soit exactement celle qui est prévue au sortir de ces débats ne finissait pas par donner l'impression d'avoir voulu donner la leçon. Alors qu'en fait vous aurez fait en sorte que le débat n'ait pas lieu, donc les leçons de politesse et les leçons de maintien, on va les mettre de côté et ce qui nous intéresse et des analyses de fond et c'est ce qu'attendent les Français, qui eux aussi dans les cortèges respecte les parcours qu'on leur donne sont très bien élevé, ça veut dire bonjour madame au revoir madame et veulent surtout savoir si oui ou non on va passer à 64 ans. Alors la parole est à madame Lubin. Oui merci madame la présidente, moi après l'intervention de notre collègue j'ai j'ai juste une question à formuler. Tout le monde sait, tout le monde sait que vous êtes très majoritaire ici et que vous êtes très très d'accord avec la route la la réforme qui est proposée par ce gouvernement. Tout le monde sait que vous avez négocié avec le gouvernement pour que la réforme qui sortira. De ce, de cet hémicycle, que si elle est votée soit tout à fait conforme à ce que vous voulez. Alors ma question est simple, qu'attendez-vous de nous. Que nous ne jouions pas notre rôle d'opposant rien et je l'ai bien entendu. Que nous ne jugeons pas notre rôle d'opposants et d'élus du peuple et c'est-à-dire que nous fermions définitivement notre bouche au prétexte que nous sommes minoritaires et que vous avez déjà tout négocier, c'est ça votre conception du débat républicain.

mes collègues je partage évidemment les propos qui ont été tenus, se sont exprimés à à l'endroit de nos collègues LR, ils l'ont fait. Dans le respect du du du à chacun. Dans le respect des formes. Et ils ont effectivement évoqué le le silence. Assourdissant qui est le leur, par rapport à la défense de de ce texte qu'il porte en réalité. Je m'étonne également. Fortement. Du si l'ANC du même si ANC de nos collègues RDPI. Qui sont quand même. Partie prenante et oh combien. De ce que contient ce texte. Voilà je crois qu'il y en a pas. Parmi eux, qui a pris la parole

Voilà et donc plus encore nos nos compatriotes ont besoin, ils nous écoutent, ils nous écoutent. Et je pense que jusqu'ici. En tout cas pour le groupe, les groupes de gauche. Dont je fais partie. Nous avons été à la hauteur des enjeux du respect des institutions et plus encore du respect des Français. vous, vous l'attendiez chers collègues de gauche et je prends donc la parole juste pour vous dire, je pense que vous nous reprochez en tout cas la majorité sénatoriale et à la majorité présidentielle. Vous nous reprochez de ne pas prendre la parole pour défendre nos amendements pour défendre article enfin pardonnez-moi, on est à l'article liminaire. pardonnez-moi aussi de ne pas forcément rebondir sur les lourdeurs, que vous avez à chaque fois répété c'est-à-dire l'Arctique préliminaire enfin vous lui avez fait trois fois de suite, donc effectivement je pense que ça ne fait rire que vous. Mais en l'occurrence, je pense que vous êtes assumer, assumer une obstruction raisonnable par rapport à celle de l'Assemblée nationale où effectivement il y avait 20.000 amendements, là on est un peu moins, un peu moins de 5000 mais assumer dans une obstruction sur nos débats parlementaires assumer le fait que vous ne voulez pas. pardonnez-moi, mais moi en l'occurrence, je vous ai écouté quand vous jure liés à chaque fois vous amendements donc effectivement assumer des dans une obstruction par rapport à vos amendements on, on voit que sur la des amendements de suppression alors que vous avez l'habitude généralement de groupés. Au sein du même groupe. Un amendement de suppression. Vous faites 62 amendements de suppression pour un article pardonnez-moi mais si c'est pas de l'obstruction c'est quoi et quand on a à chaque habitant amendements de suppression, les mêmes explications de vote qui ont été repris et tout c'est exactement la même chose. Pardonnez-moi mais. Assumer simplement d'être dans l'obstruction. Vous voulez qu'on ait le débat sur les 64 ans. Vous voulez qu'on ait le débat sur les régimes spéciaux hé bien avançons continuons travaillant sur les choses inscrites c'est ça aujourd'hui que les Français veulent de nous c'est pas l'obstruction qui a été celle qui a été organisée à l'Assemblée nationale, ils veulent de nous qu'on puisse les représenter, il veut de nous, qu'on puisse voter et faire à améliorer ce texte et pas l'attitude que vous avez aujourd'hui. Merci la parole est à madame Trix compta. Madame la présidente. Je suis très surprise de l'accusation d'obstruction parce que moi l'obstruction que je vis, c'est cette réforme des retraites dans le PLF. Parce que de nombreux amendements 1000 amendements pratiquement que nous avions proposé pour réparer des injustices parfois anciennes et qui. Entraient dans le cadre d'une réforme des retraites, ces amendements ont été rejetés, donc nous ne pouvons pas avoir un véritable débat débat sur ce projet de réforme des retraites à cause de la méthode choisie donc l'obstruction n'est pas de notre fait, mais au contraire du fait du choix de cette méthode. Cette méthode est injuste et en réalité. Quel est l'objectif de cette réforme. C'est travailler plus. Le travailler plus. Et gagner moi travailler plus longtemps pour financer d'autres choses. Que le gouvernement souhaite financer et sur ce, travailler plus, on voit bien que la majorité présidentielle et. Le, la droite se retrouve. Donc, travailler plus pour financer le déficit que l'État creuse lui-même. Je crois qu'il y avait d'autres solutions. La taxation des superprofits. La lutte contre l'optimisation fiscale. C'est quand même plusieurs plusieurs dizaines de milliards par an. Il n'y a pas besoin de faire travaille plus, ce qui déjà depuis très longtemps travaille beaucoup plus que les autres. Donc, cette réforme est vraiment injuste. Le gouvernement mise sur cette réforme pour améliorer la croissance mais on sait très bien les études macro-économique le montre que ce ne sera pas le cas, qu'il y aura une hausse du chômage, du RSA et encore davantage de personnes en grande difficulté. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Tissot. Merci madame la présidente, messieurs les Ministres, chers collègues. Je vais m'adresser à vous qui nous dites. Que nous faisons de l'obstruction mais. Finalement, croyez-vous que ce soir, vendredi soir, 23h 23, nous sommes nombreux à être finalement heureux d'être ici. Content d'être ici non. Nous sommes là parce que nous avons un mandat. Nous avons un mandat de nos électeurs qui nous ont demandé de débattre et de défendre des idées et c'est ce que nous faisons simplement moi ce soir. Personnellement, je préfère être auprès de mes enfants. Vraiment, ce soir, particulièrement particulièrement. Laissez-moi vous dire quand même aussi que moi, j'aimerais vous entendre chers collègues de la majorité sénatoriale. J'aimerais vous entendre parce qu'en fait nous allons bientôt rentrer dans une période électorale et, si vous ne vous exprimez pas ici clairement individuellement, vous allez pouvoir vous cachez derrière le propos. Ah mais moi j'ai rien dit, j'ai pas dit que j'étais pour l'allongement de la, de l'âge de la retraite que moi j'étais pas là que je ne suis pas favorable ou je ne tenais pas le discours de de de l'éloge de la paresse. Parce que je vous imagine finalement on on va côtoyer les mêmes personnes. Je vous vois difficilement dire à des gens qui vont vous vous vous sollicitez comme ils nous sollicitent, nous non non mais finalement toi certes à travailler dur. Mais tu vas devoir travailler 2 ans de plus vous tenir de tenir ce discours là et ça va être du coup plus simple pour vous si ce soir vous ne dites rien et si pendant si 11 jours qui arrive, vous ne dites rien il vous vous cachez derrière la parole de votre président. merci madame la présidente, je voulais faire un rappel au règlement, selon l'article 44 bis. Et rappeler que selon ce premier alinéa. Le gouvernement, les sénateurs ont le droit de présenter des amendements, des sous amendements au texte soumis à discussion devant le Sénat. Cela pour dire à notre collègue Xavier Iacovelli que nous ne sommes pas dans l'obstruction. Nous sommes dans l'exercice de notre fonction de parlementaire de sénateurs que de pouvoir présenter soumettre au débat des amendements. L'ennui, il est vrai, c'est que tous les amendements toutes les prises de parole sont, de ce côté-ci de l'hémicycle et comme mes collègues ont déjà pu le dire regrettait que de l'autre côté de l'hémicycle, bien il n'y ait pas du du répondant. On est là vraiment dans un espace où la démocratie doit s'exercer. On doit confronter nos points de vue et où nous pouvons. Échanger encore une fois et argumenté sur ce projet de loi. Alors nos amendements. Ils ont tous été défendue par celles et ceux qui l'ai porté avec des arguments et des objets qui ont été complémentaires les uns des autres et non pas contrairement à ce qui a été dit avec exactement la même prise de parole pour chacun et chacune d'entre nous, était, vous n'étiez-vous pas là pendant ce débat en tout cas c'est vrai qu'on n'a pas entendu de votre côté non plus. De prise de parole qui pouvait soutenir cette réforme et en particulier l'article liminaire qui est tellement important sur ce projet de réforme. Merci acte est donné de ce rappel au règlement, la parole à Monsieur Lemoine pour explication de vote. Il importe. De voter cet article liminaire. J'ai entendu sur certains bancs le fait que les dépenses de retraite resterait stable. J'ai le rapport du COR entre les mains. Elles vont augmenter dans un 1er temps, là encore pendant quelques années et après se stabiliser, mais elles vont se stabiliser à quel prix le corps l'écrit noir sur blanc, il le dit c'est principalement imputable à la baisse de la pension moyenne relative. Donc ça signifie, ça signifie que, effectivement, si elles sont stables, c'est parce que les les pensions de retraite progresseront moins vite que les revenus d'activité est ce qu'on veut se résoudre à ça non. Nous avons besoin d'agir, et c'est pourquoi cette réforme est présenté, c'est pourquoi elle doit être débattue. Il s'agit en rien d'être soumis à Bruxelles ou à quiconque. Au contraire, lorsqu'on est souverain. On prend souverainement la décision justement de ne pas dépendre de tel ou tel marché de telle ou telle instance. Et c'est donc un choix souverain que nous faisons justement pour ne pas avoir à à payer X % X milliards et caetera, le financement de tout cela et je dois dire que. Il est très important. Qu'effectivement ce débat. Se tienne dans des conditions. Bien sûr, de respect mutuel. Je crois d'examen au fond des amendements et je sais pas si c'est le fait que chacun. Dépose le même amendement qui va y aider. On sait très bien. Que dans nos débats. Il est possible, il est possible de croiser les regards de croiser les arguments sans forcément tous défendent le même amendement mais je dis ça pourquoi parce que vous avez peut-être vu cet après-midi. Une étude de l'IFOP croisant le regard des Français sur Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, regardez le résultat de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Il se fait ratatiner par Marine Le Pen sur.

Merci madame la présidente. Alors effectivement, j'ai entendu obstruction cordial. De la part. De la gauche. Moi je suis très choqué, mes chers collègues, je suis très choqué parce que l'obstruction. C'est simplement le droit d'amendement des parlementaires et vous devriez en être fier, et vous devriez le défendre. L'obstruction pour vous, c'est la défense de nos amendements. En disant d'un air méprisant qu'ils sont tous identiques, mais vous n'écoutez pas. Vous suivez un autre programme ce soir. Les amendements que nous présentons, qui sont des amendements de de suppressions sont tous argumenter en vous donnant des exemples concrets. L'obstruction, elle est réalisée. Par le gouvernement et cette réforme qui est unique et cette réforme que vous soutenez parce que là il y a le rassemblement des droites macroniste LR centristes tous ensemble pour s'en prend toujours aux mêmes ceux qui souffrent, ceux qui ont des carrières pénibles, les femmes ceux qui sont au chômage c'est toc vous attaquer. Mais le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait il fait les cadeaux toujours au même vous voulez quand on vous propose d'autres. D'autres possibilités des financements alternatifs. Ça n'est jamais bien l'arrêt. De des cotisations. Des exonérations de cotisations sociales 75 milliards, ça ne vous intéresse pas compte, vous faites par contre comme cadeau. La suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée, c'est près de 5 milliards d'euros. L'ISF 5 milliards d'euros, le CICE 20 milliards d'euros et la fraude fiscale. Mes chers collègues, collègues, c'est 80 à 100 milliards d'euros de cadeaux, ça veut dire 5 à 9 fois le montant prévisionnel du déficit annuel de l'assurance vieillesse. Alors quand on veut on peut, sans en prendre aux gens qui travaillent et qui nous regardent et qui sont heureux de voir des parlementaires digne de ce nom qui les défend. Si cher collègue, la parole est à madame Artigalas. Merci madame la présidente. Moi je vois aussi Dries répondre à quelques attaques qui nous ont été faites. Je voudrais répondre à Monsieur Iacovelli, On ne peut pas nous reprocher d'examiner de prendre du temps pour examiner et exposé des arguments contre cet article liminaire qui est quand même le coeur de la loi au détriment soi-disant d'autres articles le plus important c'est quand même les éléments financiers Nous avons pour chaque amendement deux minutes pour les défendre. Or, vous avez bien vu tous ceux tous les arguments financiers tous les chiffres quand nous ont permis d'amener tout ce que nous avons ce nous avons bien plus de temps pour exposer effectivement l'iniquité de cette loi et je vais vous dire, vous vous a dit que les journalistes pensent qu'on fait de l'obstruction mais nous, nous avons eu de nombreux sage de nos concitoyens qui regardent ces débats et qui sont très contents. Grâce à ce que nous disons d'apprendre des choses sur cette loi et de se rendre compte à quel point parfois les chiffres avancés par le gouvernement pour peuvent être. Ne peuvent, ne sont pas bons, et ensuite pour revenir, on a bien montré Monsieur Lemoine aussi la question, c'est la question des recettes. Nous avons eu l'occasion de vous donner plein d'arguments pour voir comment est-ce qu'on pouvait augmenter les recettes. De l'aide ce régime de retraite. Et je crois que là on est pas d'accord là-dessus, mais nous nous donnons aussi dans nos éléments une autre position, nous avons d'autres moyens pour retrouver un équilibre de cette réforme de cette. Le système de retraite. Merci, cher collègue, la parole à Monsieur Bourgi. Madame la présidente, mais mes chers collègues. J'ai entendu de qualificatifs tout à l'heure un collègue parlait d'obstruction cordial et le second a parlé d'obstruction raisonnable. Je considère que ce que nous faisons ici. Ça s'appelle tout simplement la démocratie ça s'appelle un travail d'opposition. Aujourd'hui nous sommes dans l'opposition. Hier vous l'étiez peut-être que le demain, vous le serez-vous à nouveau. Et ce que nous faisons aujourd'hui les droits que nous défendons aujourd'hui vous en bénéficierez le jour où vous serez vous aussi dans l'opposition. Tout à l'heure un collègue à comparer nos travaux avec ceux de l'Assemblée nationale. Comparaison n'est pas raison. Ici, personne n'a agressé les ministres. Personne n'a insulté les ministres et c'est très bien ainsi. Parce qu'ici au Sénat, nous avons le culte du respect des adversaires. Le culte du respect des ministres, le culte de la nuance et chacun et chacune d'entre nous s'il fort s'y emploie. Pour le reste. Le projet de loi qui nous est présenté, finalement c'est le projet de loi de la majorité sénatoriale par procuration. Le gouvernement le porte-par procuration. Vous devriez chers collègues de la majorité y trouver quelques motifs de satisfaction tend votre stratégie d'influence a réussi, vous avez réussi à influencer le gouvernement qui a repris à son compte ce que vous vouliez faire depuis tant et tant d'années. Réjouissez-vous revendiquer cette victoire symbolique et politique. Et vous, messieurs les Ministres vos chers collègues de la majorité présidentielle. Assumer le fait assumer seule cette jonction entre les deux droites. La droite sénatoriale, la droite présidentielle. Mais ni les uns ni les autres ne veulent assumer cette jonction parce que dans quelques semaines, les collègues de la majorité sénatoriale iront voir les grands électeurs et parmi les grands électeurs. Il y a des caissières. Parmi les grands électeurs et il y a des Atsem parmi les grands électeurs il y a des hommes et des femmes concernées par la pénibilité se sont à ces personnes-là que vous allez rajouter deux ans au compteur. Ah à ce commencer par les assumer ici parce que vous aurez à les assumer. Si chers. Il va être procédé. Scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. Alors le résultat, nombre de votants 342 exprimés, 341 pour, 250 contre. 91. L'article liminaire et adopté. Nous passons notre première partie trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune le 3394 madame pose mange. Merci madame la présidente. Mes chers collègues. Cet amendement est un amendement de clarté et de sincérité. Sur le fait que la réforme ici. Repose à 100% sur les travailleurs aucune contribution n'est demandée aux employeurs, à part la mise en place de cet index seniors. Donc il est fort probable qu'il finisse par disparaître après le passage au Conseil. Constitutionnel et qui de toute façon n'est pas contraignant, aucun effort n'est demandé aux aux aux revenus au au Patrimoine alors que selon l'Insee, en 2015 10 % des ménages français ont un Patrimoine Net supérieur à 534.000 euros. Et alors que les plus grandes fortunes équivaut au déficit des traites et qui pourrait alimenter le fonds de réserve des retraites. Vous avez participé à leur enrichissement. Nous sommes pour qu'il prenne la part de la, de l'effort. La somme de cette réforme donc repose sur les travailleurs à qui on impose 2 ans de plus alors que de multiples solutions existent dont l'augmentation des cotisations pour lesquels, messieurs les Ministres, 59% des Français sont favorables selon l'IFOP, contre l'allongement de 2 ans de leur durée de travail et 2 tiers des jeunes. Selon le chercheur Michaël Zemmour et le et le corps cette augmentation serait de 28 euros pour un salaire moyen d'ici 2027, sachant que ce même salaire augmenterait de 128 euros. D'ici là. Mais s'il faut éviter la perte de pouvoir d'achat des plus modestes pourrait sur lequel on pourrait se rejoindre. Alors l'augmentation des cotisations sur les hauts salaires est possible, d'autant que le c'est à lui-même recommandait la fin des baisses de cotisations pour les salaires au-dessus de 1,6 SMIC pour leur faible efficacité même leur leur nom efficacité. Merci cher collègue. Voilà. Nous passons à la présentation de l'amendement 3531 madame pensez c'est toujours vous. Merci madame la présidente. Alors le présent amendement relève du constat et du diagnostic partagé par toutes les organisations syndicales. Comme par les rapports évaluant déjà les effets de la loi de prolongation précédente 2010. Cette réforme frappe tous les travailleurs, mais encore plus les plus modestes et les femmes. Outre l'extension du sas de précarité et de pauvreté pour les seniors qui sont ni en emploi, ni en retraite, la réforme va impacter aussi la durée de retraite des plus précaires. Je rappelle que l'Insee ni INED le corps ont unanimement, constaté une stagnation des gains d'espérance de vie qui ne sont plus tirés que par la baisse de mortalité des plus de 70 ans. Je rappelle que selon l'adresse les réformes cumulée entre 2010 et 2015 ont déjà contribué à faire baisser, baisser la durée de la retraite de près de 7% entre la génération de 2050 et celle de 2080 et de façon très différenciées. Alors que la durée moyenne de la retraite était de 25 ans et demi avant la réforme Sarkozy Sarkozy. Elle est de 24. Demie aujourd'hui donc elle a diminué d'un an et devrait descendent à 23 ans en 2030 en projection avec cette réforme, c'est donc une marche tout simplement en arrière et selon les chefs chercheur Ulysse le jeu le Skins et et Julien Blasco de l'université Dauphine et Nanterre. La réforme envisagée diminuera la durée de retraite de l'ensemble de la population mais plus fortement des plus pauvres. Selon leurs études. Les 5% entre l'espérance de vie entre les 5% les plus aisés 5% les plus pauvres, c'est déjà 13 ans, selon l'Insee. Alors que l'espérance de vie en bonne santé entre Kurdes et un ouvrier et de 11% selon Lojkine. Les plus pauvres vont perdre jusqu'à 14% de la durée de leur retraite. Avec cette réforme, les mesures d'atténuation que vous proposez de cette brutalité que vous appelez mesures sociales n'y changeront malheureusement rien et a fortiori rien pour la très grande majorité des carrières longues

Oui, je réponds à ma collègue Raymond c'est moche pour lui dire que, en fait. La première partie s'intitule dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre de la Sécurité sociale pour l'exercice 2023. On sent bien que c'est une consonance normés et que ça ne peut pas être changé surtout avec des consonances politiques tels que vous les proposer. Donc c'est un avis défavorable. Merci madame le rapporteur avis du gouvernement.

C'est dommage que pour une fois que la majorité sénatoriale avait un amendement qui soient retirés avant d'être présenté, ça nous aurait permis d'en discuter mais du coup je vais parler des 2 amendement de notre collègue Raymond Poncet Monge et c'est dommage là que Vincent Delahaye, notre collègue Vincent Delahaye ne soit pas là parce que. Souvent, lorsqu'on discute du projet de loi de finances ou d'un projet de loi de finances rectificative. Ils proposent un amendement pour que le titre de la première partie ne soit plus dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre financier mais relatives aux recettes et aux déséquilibres financiers. Ils le présentent en disant qu'il faut mettre le titre de la première partie en adéquation avec la réalité. Hé bien ce que nous proposent les 2 amendements, 33, 94 et 35 31. Ces 2 mètres, certes avec un peu d'humour. Le titre de la première partie en adéquation avec la réalité. Donc je pense que nous pouvons tout à fait le voter. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Breuiller. Merci madame la présidente, messieurs les Ministres, bien évidemment je voterai l'amendement de ma collègue poncer Monge qui nomme les choses car mal les nommer. Vous savez que ça coûte toujours très cher. trouvent juste cette réforme 79% la trouvent injuste et je veux dire à mes collègues de la majorité sénatoriale que je reconnais, leur courage de défendent leur position alors que 59% de leurs électeurs trouvent cette réforme également injuste. les sondages, dans tous les sondages témoignent. 70% des Français par ailleurs trouve cette réforme pas clair, sans doute en partie en raison de la non-. Présentation de la note de synthèse du Conseil d'État. Au fond, le gouvernement continue à cacher des éléments des données financières c'est une Russe de procédure pour empêcher un débat sincère. Et ça n'est pas acceptable. Monsieur le Ministre, je vous redemande de produire aux yeux de tous nos concitoyens, cette note de synthèse du Conseil d'État. Mais. Si la parole est au président rénale Oui. Rémi Féraud l'a évoqué, mais sincèrement, moi je regrette qu'on ne peut pas discuter de l'amendement de Madame Boyer et de ses méthodes de ses collègues mais peut être quand même. A-t-on le droit de lire la première phrase sans la discuter sans la commenter la réforme des retraites, il nous est opposé ne va pas résoudre la question du financement de notre système de retraite par répartition, ni à moyen terme ni à long terme. C'est vrai que vous vous exprimez peu mais vous écrivez bien. Et. Sincèrement, on ne pourrait pas mieux démonter cette réforme qu'avec cette phrase je je crois que. Certaines d'entre vous ont une lucidité particulière et je voulais vraiment l'apprécier et vous dire simplement que, qu'est-ce qui gêne finalement. C'est que depuis 5 ans, vous. Un amendement d'appel, on le sait tous pour la retraite. On sait bien que la retraite 4 ans se fait pas par un amendement dans le PLFSS S mais vous un amendement d'appel. Ce qui est dommage c'est que vous ayez perdu 50 chers collègues pour déposer quelques amendements d'appel sur les vraies questions. C'est-à-dire. Comment on fait sur l'égalité des salaires homme/femme qui permet d'augmenter les recettes. Comment on fait pour que les seniors après vous proposez maintenant quelque chose mais il est bien tard. Ça fait 5 ans qu'en même temps que votre amendement. Vous auriez dû proposer des solutions pour augmenter les recettes, c'est là qu'on vous attendez, c'est là qu'on vous attend toujours et parce qu'on ne voit rien arriver. Bon mais voilà donc c'était un très bel amendement monsieur Retailleau vraiment vous n'avez pas été gentil de retirer cet amendement est de grande qualité. Merci, cher collègue, la parole est à Monsieur Lemoine. Merci madame la présidente, effectivement, une explication de vote sur le 33 94 de madame. Pour Monge. Parce que elle évoque une réforme qui suit au détriment des travailleuses et travailleurs pardon mais ça va être l'occasion puisque j'ai compris par Viviane Artigalas ce dans l'Aude, Pyrénées, on nous regardait on nous suis sûrement également dans l'Yonne, dans le Cher dans tous nos départements, hé bien c'est l'occasion également de mettre le projecteur peut-être sur des dispositions dont on parle moins et qui pourtant sont essentiels pour les travailleuses et les travailleurs. Je pense à l'article 9. Avec les départs anticipés. Songez que 40% des départs en retraite se feront sur cette base et se feront de façon anticipée regarde également les curseurs du CDP qui vont être ajustés qui vont être baissés, qui vont permettre de prendre plus de monde. Je pense également à l'article 13 sur la retraite progressive. La retraite progressive, elle existe pour l'instant seulement pour certaines catégories de personnes le secteur public n'y a pas droit. Hé bien, écoutez, le fait de pouvoir à partir de 60 ou 62 ans. Travailler à 60% de son temps seulement et puis de déclencher une partie de ses droits à retraite et ben je trouve que c'est plutôt vertueux. Eh bien c'est l'occasion de le redire et donc de dire que cet amendement effectivement ne mérite pas d'être voté ça sera un vote contre. Pour ma part. Merci cher collègue Madame Jasmin, vous avez la parole. Merci madame la présidente. Bien, je suis vraiment séduite par l'amendement de notre collègue Valérie Boyer. Parce qu'en fait ça va dans le sens de ce que je disais hier. Je parlais de la démographie. Je parlais de la démographie et de la situation des femmes. Il y a justement, il y a une quinzaine de jours déjà lors des questions au gouvernement, mais là je trouve que Valérie Boyer a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment dommage qu'elle n'ait pas pu défendre parce que je l'aurais probablement voter. Parce qu'elle pas effectivement la situation des femmes mais ont des femmes qui sont en âge de procréer qui voudraient faire des enfants et travailler aussi et hier encore je le diesel. J'ai eu seulement 4 minutes mais j'ai parlé de la démographie. J'ai parlé de la situation des femmes et de la précarité également merci Valérie Boyer pour ce que vous avez fait malheureusement. Je ne suis pas d'accord avec le fait que vous ayez évidemment. Arrêté dans votre belle lancée parce que vous ne l'avez pas présenté mais franchement les arguments sont très très bons et franchement j'aurais pu faire le même. Merci. Merci, cher collègue, la parole est à Madame Lienemann. J'ai réagi après l'intervention de notre collègue Lemoine qui a bien du courage. Pour essayer de trouver quelques éléments. Qui comme une rustine dans un système de, en train de se se d'être détérioré pourrait rattraper la donne. Il nous a dit tout à l'heure et en cela je rejoins l'amendement de Madame. Ponce. Il nous a dit tout à l'heure vous allez vous avez baissé les retraites avec la loi Touraine enfin vous, certains ont baissé les retraites avec la loi Touraine les Avec notre réforme ça va pas être le cas. D'un manque de chance, ça va être pire. C'est-à-dire le niveau des retraites. Va considérablement baissé et en tout cas si on compare le ratio entre les retraites et les salaires. je rappelle que le et. Pourquoi, parce que plus vous accélérer. La réforme Touraine. Plus vous mettez une accélération sur la baisse des retraites. Ce qui va avoir lieu. C'est que. La projection 1% c'est-à-dire celle du corps la pension moyenne passerait de 50% du salaire moyen en 2021 à 42% en 2050. On est vous votre réforme accentue encore ce phénomène, il faut le dire aux Français oui ses comptes les travailleurs non seulement ils vont travailler plus mais leur retraite va considérablement baissé et d'ailleurs. Puisque vous nous donnez toujours les exemples étrangers. Je vous rappelle qu'en Allemagne. Le taux de retraite. Ne dépense même à la fin du temps de cotisation ne dépense jamais 50% des revenus. Des actifs. Et vous avez un pays où le nombre de retraités pauvres ne cesse de s'accroître. Alors votre modèle. Certes, la France est généreuse, mais surtout la France elle est respectueuse de la dignité humaine et faire que les retraités. Moi je suis un peu l'allégement de la pauvreté parole pas républicain. La parole est à madame. Mon. Oui alors merci notre collègue le Moine de de prendre la parole. Alors effectivement, il parle de l'élargissement des départs anticipés pour carrière longue. Et d'ailleurs de la création de des super-carrières longues.

Tout comme il aurait pu parler que ils vont revalorisé de 0, 0 c'est important à 100 les minima contributif mais sur ces 3 points. Il oublie de préciser une chose. Contre 2 ans de travail de plus enfin. Les la fameuse départs anticipés pour carrière longue qui avait été obtenu à 60 ans qu'on est passé à 62 ans. passe à 62 ans qu'on passe à 64 et vous envisagez peut-être dans 5 ans, de passer à 64, on passera 66 donc. Vraiment à chaque fois. Dites nous revalorisons les minima contributif de 0 beaucoup, 0 à 100, contre 2 ans de travail en plus. Nous favorisons la retraite progressive mais qu'à partir de 62 ans. Désormais nous. Enfin. Favoriseront les départs anticipés pour carrière longue mais là aussi, 2 ans plus tard. Y'où Monsieur Savary. Monsieur le rapporteur. Vous avez la parole. Oui merci madame la présidente. Simplement je remercie Madame Lienemann qui connaît bien ces dispositifs et de qui a bien exprimé la réalité de la situation, elle a bien dit. Le fait d'étendre la réforme Touraine arrive à DC les pensions. C'est bien ça l'équilibre et effectivement on sait très bien que la réforme Touraine en allongeant la durée de cotisation sans bouger à l'âge fait que les retraites moyennes vont baisser de 300 euros dans quelques années, le fait de décaler l'âge évite de partir avec une décote et c'est la raison pour laquelle ça augmente les pensions de retraite. En plus vous avez des années supplémentaires qui permettent, qui permettent effectivement de faire en sorte que les retraités bénéficient d'une meilleure retraite. C'est la raison pour laquelle nous expliquons depuis 4 ans qu'il faut être attentif à ces 2 piliers qui constituent notre système de retraite. Le pilier de la durée qui protège ceux qui commencent tôt. Le pilier de l'âge qui protège ceux qui commence tard et si vous ne jouez pas l'articulation avec les deux, vous avez un système compte tenu de la démographie, compte tenu du nombre d'entrants qui diminue de plus en plus compte tenu de la longévité qui fait que la durée de retraite augmente de plus en plus qui va à au déséquilibre le plus complet. Si nous ne prenons pas nos responsabilités. Aujourd'hui,

nos enfants travailleront pas 43 ans. Ils travailleront 45 à 46 ans, ce sera le seul mouais façon d'équilibrer le dispositif. Alors, mes chers collègues, nous aurons l'occasion de discuter de cela pendant plusieurs jours et c'est la raison pour laquelle face à cette demande supplémentaire d'un effort les. This. Le Sénat va vous proposer des mesures de justice sociale qu'on. Si monsieur le rapporteur. La parole est à monsieur Marie. Merci madame la présidente. Monsieur le rapporteur. Vous voulez nous expliquer que vous allez nous faire des propositions. Et. Que. Dans l'état actuel de la réforme. Les retraités gagnerait plus. J'ai vous parlez. De quelques-uns de nos concitoyens. Quelques millions de nos concitoyens. Ceux qui. Aujourd'hui ont. 60 ans et qui pour un tiers d'entre eux. Ne sont ni en emploi, ni à la retraite mais. Soit au chômage, soit au Revenu de Solidarité Active. Soit en invalidité soit en congé de maladie. À 61 ans ils sont 61% à être dans cette situation. À 62 ans ils sont 73. 6 % à être dans cette situation. Alors imaginez combien ils seront à 63 ans et combien ils seront à 64 ans et si pour eux le fait d'attendre encore 2 ans pour sortir de la précarité est véritablement une avancée sociale. Merci, cher collègue, la parole est à madame Lubin. Il est une constante dans toutes les réformes des retraites et qui ont été faites après celle qui a amené la retraite à 60 ans qu'elles ont toutes baissé à terme le niveau des pensions, la pire à mes yeux, a été celle de 93. Qui a fait que l'on a calculé la retraite du privé sur les 25 meilleures années. Au lieu de la calculée sur les 10 meilleures années, ça a été un cataclysme pour beaucoup de salariés du privé et que l'on a indexé ses l'évolution de ces retraites sur les prix, c'est ça qui a été catastrophique pour les salariés du privé et les autres. Réformes qui ont suivi n'ont pas apporté non plus d'amélioration. La réforme Touraine tout le monde dit tape dessus Je ne renie pas quand même tout à fait ce que je suis et ce que j'ai. À un moment soutenu la réforme Touraine. Quand elle a été faite la projection immédiate. Je rappelle quand même qu'on était vraiment sortir on était encore pas sortie d'ailleurs de ces fameuses années de de crise. Elle a été faite à un moment où la projection de déficit était de 30 milliards d'euros. Aujourd'hui, on est toujours pas en déficit hein je le rappelle quand même. Est certes elle à allonger la durée du travail, c'est vrai mais elle a maintenu 62 ans. D'aucuns diront c'est de l'hypocrisie. Mais moi je, non non, chers collègues. Tous les Français ne font pas des études supérieures, très longue, il y a encore beaucoup de gens et il y en aura toujours qui commenceront à travailler à 18, 19 et 20 ans et ceux-là, je suis désolé mais il faut les protéger, là on est en train de faire comme si tout le monde commençait entrer dans la vie active à 25 ans. Mais non c'est pas vrai il y a pas de catégorie de Français il y a une seule catégorie de Français et certains il faut les protéger plus que d'autres et on aura l'occasion d'en reparler j'aurais encore plein d'arguments. Merci cher collègue. Je vais mettre aux voix l'amendement 3394 car. Monsieur Lurel. Vous souhaitez la parole pour explication de vote. Oui merci madame la présidente. Notre collègue ça varie vient de nous expliquer qu'il y a deux variables. Je n'ose pas dire. De paramètres ce que c'est une réforme paramétrique. Vous ne tenez compte pas compte des verts des choses qui évoluent de variable la durée et et l'âge. Ce raisonnement ne peut tenir que si vous ignorez l'environnement général. Le système lui-même parce que dans votre conception de. Du régime par répartition. Seuls les salariés. Cotisent et doivent équilibrer leurs Vous refusez de comprendre que le système par répartition qui est déjà financé à 54% par les cotisations, le reste par subventions, dotations et que sais-je encore, que ce système-là est équilibré qui libérables et qu'il tient la route dans la trajectoire si vous tenez ce raisonnement effectivement c'est de l'impro pied de l'année entropie pour parler comme les physiciens forcément il y a une dégradation qui va s'opérer, mais si vous l'ouvrez et que vous dites, je peux faire payer plus de CSG j'ai plus de dividendes plus de superprofits. Le système est parfaitement pérenne able. Et il est parfaitement durable. Si je mets maintenant aux voix l'amendement 3394 qui a reçu 2 avis favorable de la commission et du gouvernement.

Alors sur l'amendement 3530. Tiens je suis saisi d'une demande de scrutin public par le groupe écologiste solidarité et territoires. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable. Avis du Gouvernement défavorable à il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement, le scrutin est ouvert.

Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. 91 contre 251. L'amendement n'est pas adopté. Non là. C'est bon article additionnel avant l'article 1er, l'amendement 4473. Qui le présente. Madame pour ce.

L'argument irréfutable brandie par tous les membres du gouvernement repose tantôt sur les registres. Il y a un déséquilibre insurmontable entre actifs et retraités, on vit plus longtemps on doit travailler plus longtemps à chaque occasion quand cela ne suffit plus, il suffirait pour le ministre de dire que nous sommes les seuls à résister aux grands phénomènes structurant du continent européen que tous les pays qui nous entourent aurait réformer leur système de retraite en somme que les Gaulois réfractaires, s'opposerait à la raison. Ces mêmes arguments justifie la brutalité de la réforme. Un des soutiens d'Emmanuel Macron de la première heure Elie Cohen, cité par Public Sénat explique sur un plateau de télévision, brandissant la carte des âges légaux de départ en Europe que n'importe qui peut constater que ces chiffres montrent que la France est une espèce d'oasis au milieu des pays européens et justifie la nécessité de la réforme, par un déficit démographique, l'âge moyen de départ à la retraite et selon la page 51 du rapport du COR de 63 années en France. Un an de plus pour l'âge légal. L'OCDE estime elle l'âge de départ moyen de la France à 64. Contre une moyenne de 63 9 en Europe. Un travailleur français travaillent donc en moyenne sur sa vie plus longtemps qu'travailleurs européens et si ça n'était pas le cas, serait-ce une condition suffisante pour faire passer en force cette réforme injuste sans aucune contribution du capital. Comment ne pas repenser aux propos tenus le 4 décembre 2020 par le ministre de l'économie Bruno Lemaire qui a défendu sa volonté de continuer la réforme des retraites en affirmant que sur l'ensemble de la durée de vie, collectivement, nous ne travaillons pas suffisamment. Un ministre qui avait passé la première année de la crise sanitaire a demandé aux Français d'applaudir les premiers de corvée.

C'est monsieur Guy qui a la parole. Ce qu'on fait. Merci madame la présidente. Messieurs les ministres, mes chers collègues. Oui, nous demandons d'avoir un rapport, je sais que le Sénat. N'apprécie guère, enfin ça dépend lesquels. Parce que il y a beaucoup d'éléments qui sont données sur la table mais on va pas au bout des débats par exemple, on nous dit, comme l'a dit ma collègue Katia pour se. 62 ans c'est une moyenne basse et tous les autres sont à 65 voire 67 ans sauf que déjà dans notre droit français. Il existe de bornes aujourd'hui 62 ans. Pour l'âge légal mais 67 ans comme les autres pour ne pas avoir la suppression de la décote. Donc il faut comparer ce qui est comparable. Parce que dans d'autres pays européens, il n'y a pas ces de bornes 2ème question on veut comparer ce qui n'est pas comparable. Nous sommes un des rares à avoir un système par répartition. Tous les autres sont par un système de par capitalisation. D'ailleurs, l'ancien directeur de la Sécurité sociale suédoise. Qui a effectué. Cette réforme il y a 20 ans nous implorent. De ne pas le faire. Parce que il implore Emmanuel Macron de ne pas le faire parce qu'il a vu les dégâts que ça faisait sur les retraités en Suède ou alors il y a un agenda caché et ce qu'ils disent la main sur le coeur qui défendent le système par répartition veulent passer à la capitalisation d'ailleurs euros dis que nous nous rappelons de 2019 et enfin dernière chose qu'il nous faudrait approfondir le nombre de retraités pauvres. Par exemple on se compare beaucoup avec l'Allemagne. Ah oui quand on est passé de 65 à 67 ans la projection c'est qu'on va passer de 15 à 21%. Dorothée très pauvre comparé à la France ou et c'est déjà trop. Nous sommes à 10% et donc nous pensons qu'il faut un rapport pour approfondir, toutes ces questions et que nous puissions évidemment légiférer dans des bonnes conditions. Je vous remercie. Merci monsieur Gay la parole à monsieur le comte pour explication de vote.

La chance d'avoir cette demande de rapport. Validé. D'abord parce que effectivement c'est important de comparer. Nous voyons un certain nombre de pays qui ont mis en place des systèmes de capitalisation et qui sont revenus en arrière et qui sont revenus en arrière en constatant que dès lors qu'ils avaient un déficit budgétaire les régimes par capitalisation. Aggraver le déficit budgétaire et ne servait pas l'intérêt général et sont revenus en arrière et énormément de pays de l'Union européenne ont fait cette observation. Deuxièmement, il est important de comparer parce que les systèmes dans l'Union européenne sont. Harmonisées au niveau de l'Union européenne. Sauf que sauf que bien entendu l'harmonisation se fait pas nécessairement pour le bien des personnes qui sont en mobilité et c'est vrai que dans votre rapport, si vous voulez que je voulais le, le sous-amendé, il y a aussi besoin de savoir comment les personnes qui sont en mobilité peuvent effectivement bénéficier en particulier de. D'une bonne continuité de leur carrière. Je pense à 2 aspects. Le premier aspect, c'est la capacité d'avoir le taux de leur retraite pour la retraite française qui prend en compte l'ensemble des parties de carrière qui ont été faites à l'international. Le régime européen le permet. Sauf que d'un pays à l'autre, la manière de compter les choses n'est pas le même et c'est important que ce soit inscrit dans un rapport pour quand on harmonise parfois harmoniser par le haut, en s'inspirant des bons exemples et pas nécessairement des mauvais et la 2ème chose c'est que effectivement quand on a une partie de carrière à l'internationale et en particulier en Europe, la question qui a été évoqué par Marine Le Lienemann tout à l'heure des 25 meilleures années. Si vous faites la moitié de votre carrière en France et d'autres moyens de votre carrière en Allemagne. Et qu'on vous pose la question, que le 25 meilleures années en France. Eh bah c'est toutes vos années.

Merci madame la présidente. Alors moi je remercie Katia pour se polie pour avoir dénoncé un autre mensonge, celui qui dit qui nous dit, on vit plus longtemps. Il faut donc travailler plus longtemps. C'est ce que disait monsieur Sarkozy en 2010 et ils disait même. Il aime beaucoup la règle de Monsieur Sarkozy pour les 10 pour les profits, dit un tiers pour les travailleurs, un tiers pour le capital, un tiers pour l'investissement et pour l'espérance de vie il disait 2 tiers pour le travail et un tiers pour la retraite. De fait, depuis sa sa réforme, 2010, on a mangé.

diminué d'un an donc hein on a boulotter les de 100% des des gains d'espérance de vie et on a pris sur la durée de la retraite et votre réforme c'est de nouveau prendre sur la durée de la retraite, je l'ai dit tout à l'heure les projections sont sont scientifiquement démontré. Plus d'un an à la durée de la retraite, donc c'est effectivement un grand mensonge et merci. À cet amendement du groupe communiste d'en parler. Merci la parole est au président. juste un mot pour. Saluer cette demande de rapport. Parce que. Qu'est ce qu'elle veut faire finalement cette demande. c'est d'abord peut être faire en sorte qu'il y ait une vraie étude d'impact qui ne soit proposé de cette réforme parce que quand même quand on regarde. L'importance de ce sujet, je parle pas uniquement de l'importance financière, je parle de l'importance sociétale et que l'on voit comment ça a été traité en terme d'étude d'impact, c'est d'une pauvreté affligeante et que donc effectivement avoir une vision. Européenne un peu solide sur ces sujets là c'était quand même quelque chose d'absolument nécessaire pour, pour démarrer, donc moi je ne vois vraiment que du positif. Dire qu'on parle toujours des choses qui sont difficiles, on vous dit par exemple dans certains pays nordiques. Les gens vont jusqu'à 65 ans sans problème. Voire plus mais en même temps si on en fait on a eu des études comme ça qui nous ont été transmises. Quand on regarde la qualité de vie au travail dans ces pays et en France on est avant-dernier en Europe. C'est-à-dire que la qualité de vie au travail, âgée elle est considérée comme. Très mauvaise en France quand effectivement dans un pays, on se sent bien au travail et qui a une organisation du travail qui est fait autour de l'idée que l'on peut poursuivre longtemps une carrière au sein d'une entreprise par exemple, hé bien de toute évidence on accepte plus facilement des, des contraintes liées à l'âge de départ à la retraite mais c'est tout ça qu'il faut arriver à mesurer avant d'arriver sur quoi que ce soit qui soit de nature financière. Donc évidemment, je suis très favorable à cet amendement. Merci cher collègue. La parole est à Madame Lienemann. Oui, ce rapport sur la situation notamment comparative en réalité du niveau des retraites en Europe, extrêmement importante. Pourquoi, parce qu'on commence à raconter n'importe quoi. Et la plupart du temps, toujours pour dévaloriser le système français qui serait coûteux de la gabegie pas efficace économiquement et L'Italie avait modifié son âge de retraite avec monsieur Mario Monti. Malgré son âge légal à 67 ans. La part de dépenses des retraites dans le PIB n'a fait que s'accroître. Et d'ailleurs c'était tellement insupportable. Que le gouvernement italien a dû revenir en réalité à pouvoir partir à 62 ans avec 41 annuités cotisées. Pour une raison simple, c'est que c'était tellement un affaiblissement du niveau de retraite et un mécontentement social que ils ont dû reculer. En Allemagne, les comparaisons sont extrêmement édifiante. Le niveau des retraites est particulièrement bas. Et le nombre de retraités de plus de 69 ans qui travaille est considérable. Je veux bien que ce soit le fin du fin de la compétitivité mondiale. Mais très honnêtement je j'd'ailleurs la plupart du temps ce n'est pas dans les secteurs de forte compétitivité que ces emplois sont trouvés car on le sait aussi. Plus nos concitoyens sont âgés, plus ils ont des problèmes de santé, des problèmes d'adaptation aux évolutions technologiques et toutes les formations que vous voulez faire au dernier moment vu les gap technologique que nous connaissons sont inopérantes. Donc oui, nous avons besoin de ces comparaisons. Et contrairement à ce que j'entends comme discours dominant ou le système français serait toujours le même le

Merci madame la présidente. D'abord je dois dire que je suis fier si notre pays a le système de retraite le plus généreux. Vous savez que j'aime beaucoup ma ville d'Arcueil. Lorsque j'ai été élu maire, j'ai été rechercher à l'intérieur de nos archives il y a 70 ans, le CCAS s'appelait le bureau d'aide aux vieux travailleurs. Eh bien heureusement, grâce aux retraites grâce aux progrès sociaux aujourd'hui le CCAS ne s'appelle plus le bureau d'aide aux vieux travailleurs malheureusement il s'intéresse beaucoup à la jeunesse aux travailleurs précaires et à toutes les gens qui sont malmenés par notre société. Ceux qui ont des carrières hachées et tous les travailleurs pauvres qui seront pénalisés par votre retraite je soutiens évidemment cette demande d'étude d'impact. C'est toujours intéressant de se comparer, en comparant la totalité des éléments y compris le taux de pauvreté mais aussi éventuellement la richesse de la vie associative permis par le système de retraite français excusez-moi chers collègues du groupe CRCE je soutiens pleinement votre demande. Mais avant d'avoir votre rapport j'aimerais avoir le rapport. Du Conseil d'État. Celui-là il est écrit. Et pourquoi le cacheton aux parlementaires et pourquoi le cacheton aux Français parce qu'il dit que le véhicule utilisé va rendre inconstitutionnelle. Tout ce qui va atténuer la dureté de la réforme que vous faites et ça c'est aussi ce qui va nous empêcher de déposer des amendements d'amélioration de toutes ces considérations. Donc ça n'est pas une demande pour faire des effets de scène je redemande, Monsieur le Ministre, que vous nous donniez ce rapport et je termine en vous remerciant, messieurs les Ministres parce que la concision de vos réponses ne nous noie pas sous des monceaux de chiffres ou de d'arguments techniques incompréhensibles, vraiment merci pour votre concision. moi je voulais juste te dire qu'effectivement c'est intéressant de faire des comparaisons parce que. D'avoir au moins des éléments scientifiques parce qu'on entend beaucoup de choses. Qui sont souvent fantasmé et puis on entend des choses. Qui auraient tendance à dire que ben finalement. Comme on a mieux que tout le monde, il faut qu'on fasse moins bien. Et ça c'est un raisonnement que j'ai du mal à comprendre, j'allais dire nous sommes censés partir plus tôt que les autres. Enfin je vais pas refaire les raisonnements qui ont déjà été fait alors que nous sommes censés avoir les retraites meilleur que les autres nous sommes censés plein plein de choses et donc finalement la morale de tout ça. C'est qu'il faut qu'on légifère pour avoir moins. J'avoue que je ne comprends pas bien. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Marie. Merci madame la présidente. Cet. Amendement du groupe CRCE demandant un rapport au gouvernement. Et très intéressant. Ça a été. Dit par d'autres avant moi. Il est clair que. L'approche européenne pour déterminer les meilleures solutions est une approche extrêmement intéressante car en France. On part en général. Après l'âge légal et la moyenne aujourd'hui ses 63 ans. Dans le reste de l'Europe. Et dans beaucoup de ces pays. C'est l'inverse. On part avant l'âge légal. Avec des cotes. Et donc. La question de fond n'est pas tant celle de l'âge pivot. Mais celle. Du montant des rémunérations perçues lorsqu'on est en activité. Le montant des cotisations qui sont versées et donc in fine et le montant de la pension au moment du choix de départ et donc quand on regarde précisément les comparaisons entre pays. On constate que dans un bon nombre d'entre eux. Les Européens partent. Avant les Français. Avec des niveaux de pension équivalent voire supérieur. Parce que leur système a été conçu comme cela et donc je pense qu'effectivement il y a des leçons à en tirer. Et donc cette étude. Et ce rapport serait extrêmement utile avant que nous prenions des décisions définitives. Merci monsieur Marie. La parole est à monsieur Laurent. Monsieur le président. Merci madame la présidente. J'interviens, non pas pour en rajouter sur les arguments qui ont été donnés mais pour demander une précision au rapporteur de la commission puisqu'il puisqu'il y a pas eu d'avis motivé, on a juste eu un avis défavorable, sans aucune motivation. Alors je voudrais savoir, parce que souvent, par rapport au rapport. On les, vous les éliminer de manière un peu systématique, je voulais savoir s'il y a une règle qui a été fixée pour refuser tous les rapports qui vont être proposés par les différents bancs de l'hémicycle, puisque j'ai vu qu'il avait des amendements qui allait de proposer sur ces bancs, mais des amendements qui de rapports qui allait de proposer sur les bancs de la majorité sénatoriale, donc est-ce que vous êtes donné comme règle de refuser tous les rapports. Et si ce n'est pas le cas. Quels sont les critères. Pour en accepter certains et ont refusé d'autres et à ce moment-là, j'aimerais savoir pourquoi vous refusez celui-là s'il n'y a pas mais si c'est une règle générale. Je défendrai quand même le rapport mais ce sera un argument, s'il y a pas de règle générale, je voudrais connaître les arguments qui conduisent à refuser celui-là. Madame la rapporteure. comment dirais-je, qui n'ont pas un avis favorable. Par contre, ça n'empêche pas l'assemblée de voter favorablement sur certains rapports bon mais là pour l'instant on on est sur le premier là donc on l'a pas encore voté. Donc peut-être qu'il sera voté par l'Assemblée. Si vous êtes très persuasif.

Oui mais là si on l'a gardé René-Paul. Excuse-moi, excusez-moi parce qu'on a une conversation entre nous là. C'est vrai que vu le nombre d'amendements. On a quand même eu quelques comment dirais-je ajustements qui ont été assez. Rapide et et qui se sont faits de façon voilà très rapproché non pas expéditive. On les a tous regarder malgré le nombre croyez-moi et ça nous a pris du temps avec René-Paul mais cependant, je voudrais rappeler que les rapports au Sénat ne sont ne font guère l'objet d'un avis favorable des commissions parce qu'on sait que chaque année il en est tellement demandé mais c'est vrai il en est tellement demandée qu'il en est tellement peu qui sont finalement produit parce qu'on ne peut pas non plus imaginer. De de de demander au gouvernement de toute façon sur. Le le le rapport que vous souhaitez là sur la comparaison avec les pays européens. Je voudrais vous rappeler que dans les annexes. Vous avez un certain nombre d'éléments que vous pouvez retrouver et d'ailleurs qui sont en faux par rapport à ce que certains ont déclaré tout à l'heure on pourra. Vous le dire mais en tout cas moi je vous suggère de de de demander à Madame Lienemann qui a l'air de connaître absolument bien l'ensemble des pays européens en tout cas en terme de retraite et vous avez un rapport toute de suite produire. Je je je le propose. Merci madame la rapporteure. La parole est à monsieur sueur pour explication de vote. de vote. Aussi faire un rappel au règlement sur l'article 40 de la Constitution, en effet, j'ai écouté avec soin ce que vient dire de dire Madame la rapporteure. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas c'est que un certain nombre certains d'amendements déposés par des collègues. N'ont pas reçu un avis défavorable. Ce que vous venez d'expliquer, on comprend cela très bien. Mais ont tout simplement été frappé par l'article 40. j'ai écouté ce qu'a dit notre président de la commission des finances, notre ami Claude rénal qui s'est félicité que ce rapport que ce que l'amendement soit. Adopté au puisse puisse être adopté ne l'pas encore. Mais je ne comprends pas pourquoi un certain nombre d'amendements proposant des rapports. Sont invalidées au titre de l'article 40. Pourquoi parce que oh présuppose. Que le fait qu'il y ait ces rapports pourrait. Induire des dépenses ou des charges complémentaires pour l'État. Et ça, ça n'a pas de justification puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le rapport est un rapport n'entraîne pas de coup particulier alors maintenant. On nous dit aussi que c'est l'article 45. Mais comme je peux aussi répondre là-dessus. Si c'est l'article 45. Alors il faut m'expliquer amendement après amendement et nous pourrons peut être le dire lors des explications de vote lors lors des votes sur les articles en quoi. Ces amendements n'ont pas un rapport, même indirect avec le texte puisque je précise là je parle de l'article 45 de la Constitution. Il dit que les s'amendements sont acceptables dès lors qu'ils ont un rapport même indirect. Or la plupart de ceux

Monsieur le comte, vous avez déjà eu là. C'est. C'est un détournement de procédure. Monsieur Lurel. De mer. Si madame la présidente. Tu auras droit tout à l'heure à ton appel au au règlement. Jean-Pierre Sueur notre collègue lorsque vous avez la constitution de la Ve République qu'on l'utilise au maximum toutes ses ressources qu'on impose une loi de financement qu'on refuse l'avis du Conseil d'État que bon on l'Arctique hein, qu'est ce qui reste à un député ou un sénateur. L'arme du pauvre, l'amendement. Et une demande de rapport pour contourner cet article 40 je parle pas du 45 le. J'aime bien m'habiller. Défendu. Qu'est-ce qui nous reste, c'est demander des rapports et avant d'aller en Europe. Je reste chez moi un Guadeloupéen Martinique et c'est la même chose dans, dans tous les outre-mer français si on avait fait un rapport avant on aurait pas proposé cette loi la telle quelle sans différenciation aucune sans pour autant demander à toucher à l'unité de la République. Si on avait fait. Un rapport si on avait fait une étude d'impact, si même il y avait une fiche d'évaluation comme on on nous l'a imposée. Peut-être que ce texte là ne s'applique pas. La seule chose qui nous différencie le seuil de récupération sur succession hé bien le ministre propose de le supprimer, alors qu'il suffisait simplement de dire ça s'applique à toute la République française c'est pas 39.000 euros c'est 100.000 euros mais voilà il faut des rapports et il faut être un peu moins aveugle. Merci Monsieur Lurel monsieur le comte. Vous avez déjà eu la parole. Donc c'est un rappel au règlement, alors. C'est sûr que l'article 17 bis. Le le 17 bis. Parce que je voulais. Aussi rappeler ce que j'avais évoquée tout à l'heure nous avons a effectivement un certain nombre de demandes de rapport qui sont déclarés irrecevables. Pas au titre de la l'article 40 ou 45 mais au titre de la loi, la loi organique et de l'article L O 111 3 12 du code de la sécurité sociale. Pour quelle raison. quand je comprends ce que m'écrit la présidente de la commission des affaires sociales. C'est parce qu'un rapport n'a pas d'effet sur les comptes de la Sécurité sociale. Comme la. C'est quand même assez étonnant parce que à ce moment-là, ça veut dire que dans toute loi de finances, on ne pourra plus jamais demandé aucun rapport si cette. Cette explication est fait, moi je suis quand même étonné de voir par exemple un amendement que je dépose le 2333 l'irrecevabilité et déclaré parce que alors c'est un article et on me le la la président de la commission du personnel à me dit cet article, cet amendement qui prévoit la remise d'un rapport sur les modalités de calcul des pensions. C'est quand même au coeur du sujet. Ne porte pas sur l'application d'une loi de financement de la Sécurité sociale. Il est donc irrecevable en application de l'article dans l'article L O 111 3 12 du code de la sécurité sociale. Alors je veux bien qu'ils n'aient pas d'influence directe sur les comptes de la Sécurité sociale puisque c'est un rapport qui ne coûte rien, qu'il ne rapporte rien mais ça relève du contrôle de du Parlement et cette multiplication de l'Arctique de de de

de son travail de parlementaire sur un sujet particulièrement lourd à partir du moment où effectivement si on propose des modifications qui coûte, on ait attrapé de l'article 40, il est quand même logique de demander un certain nombre d'études d'impact sur les choses que nous voulons voir modifier. Voilà et c'est la raison pour laquelle je pense qu'avec ce type d'application. Hé bien, madame la présidente de la commission des affaires sociales fragilise l'appliquer le l'examen de l'ensemble. Les Tigers merci. Il me semble que même la présidente avait déjà expliqué plus tôt dans la séance. La façon dont elle avait appliqué les y'recevabilité au niveau de la commission et qu'elle s'en était déjà exprimé. Madame Jasmin. Oui merci madame la présidente, je voudrais justement aller dans le sens de ce qui a été dit par Victor et Lionel mais dans le sens également de la demande de Madame Assassi. Si. L'étude n'est pas que l'avait été fait avec les données de la CNAV. La CNAV, qui a été cité hier par monsieur Retailleau mais aussi dans mon intervention j'en ai parlé, hé bien si les données avaient été suffisamment exploité. Eh bien nous aurons vu justement les incidences statistiques mais aussi réel. Sur notre population des le le chèque que les territoires d'outre-mer et là, ça n'a pas été fait donc on là je disais qu'il n'y avait pas eu d'étude d'impact préalable et là je crois que si on fait un travail sérieux, ce serait important d'exploiter les données réelles de la CNAV, qui sont connus, qui sont on peut exploiter à tout moment. Eh bien je crois que ça facilite les notre travail de ce soir. Si, alors je pense qu'on a épuisé les paroles. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe CRCE sur l'amendement 4473 je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable. L'avis du Gouvernement défavorable. Il fait procéder au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement, le scrutin est ouvert.

contre 251. L'amendement. N'est pas adopté. Mes chers collègues, je vais lever la séance, nous avons examiné. 77 amendements au cours de la journée. Il en reste 3657 à examiner sur ce texte. Prochaine séance samedi 4 mars à 9h 35 pour la suite du projet de loi de financement rectificative de de la sécurité sociale pour 2023. La séance est levée.